Je souhaite l'exprimer également dans cet hémicycle. Le malaise des policiers, c'est celui d'agents qui craignent pour leur vie, laquelle ne représente rien pour les voyous, ceux-là mêmes qui tentent de les brûler vifs à Viry-Châtillon, leur tirent dessus à bout portant à Avignon, leur jettent des parpaings à la figure n'importe où. où. C'est aussi le doute des policiers, des gendarmes, qui s'interrogent de plus en plus sur le sens de leur engagement. On peut en effet tourner le problème dans tous les sens- recruter plus, acheter plus de voitures, verser des primes, créer des observatoires -, rien n'y fait. Le problème, c'est qu'à peine arrêtés les délinquants sont déjà relâchés dans la nature. Que ressent le policier qui vient d'interpeller un délinquant en flagrant délit quand celui-ci est libéré dans les heures qui suivent, qu'il passera pour un caïd auprès de ses copains, alors que lui est encore occupé à remplir la paperasserie de l'interpellation ? Et que pense le concierge lorsqu'il retrouve le même individu, arrogant et menaçant, dans la cage d'escalier, quelques heures plus tard ? À cet agent, à ce concierge, aux victimes, on dira que l'on n'a pas jugé utile de le placer en garde à vue ou que le délinquant a refusé sa comparution immédiate, mais qu'il y aura bien un rappel à la loi ou de la prison avec sursis dans quelques mois ou trimestres. Ces réponses quotidiennes et répétitives sont inaudibles. Elles engendrent le sentiment d'impuissance et la conviction d'impunité elles font naître le désarroi et l'humiliation des honnêtes gens. L'autorité de l'État ne se décrète pas : elle se manifeste et elle s'impose. Mes questions, monsieur le Premier ministre, sont donc simples : quels actes forts le Gouvernement entend-il prendre pour mieux protéger ses agents ? Doit-on modifier notre échelle des peines afin que la sanction visible et immédiate devienne désormais la règle ? La parole

Permettez-moi d'exprimer un désaccord : nous aurons créé, au cours de ce quinquennat, 10 000 postes supplémentaires en net sur les forces de sécurité intérieure, est quand même mieux que d'en avoir supprimés, comme cela a pu être le cas, je le rappelle, par le passé. Dont acte

pas. Pour faire face à la vague de violence contre ces mêmes forces de sécurité, et, au-delà, contre les citoyens de ce pays, il faut aussi que la réponse pénale suive.

pareil pour l'ensemble du service public de la justice. Le problème vient de très loin. Il nous faut restaurer ce service public et réparer tous les maillons qui font défaut. J'en citerai quelques-uns.

Aussi, dans le cadre du Beauvau de la sécurité, nous allons la restaurer, y affecter davantage d'effectifs, mieux les former, mieux les qualifier, pour que les affaires arrivent en état d'être mieux jugées par l'autorité judiciaire.

pour mettre au service de la numérisation de toutes nos procédures les moyens qu'il faut. J'ajoute qu'évidemment la représentation nationale sera saisie

dans les zones d'éducation prioritaire, c'est aussi lutter contre l'insécurité. Nous devons agir sur tous les registres. L'État est ferme ; l'État est décidé : il ne laissera personne abîmer la République

le Conseil de sécurité des Nations unies, verrouillé par les États-Unis, s'est réuni trois fois, sans résultat. La liste des morts et des blessés s'allonge de part et d'autre. Cependant, l'immensité majorité des car la disproportion de l'usage de la force est évidente. Monsieur le Premier ministre, hier, à l'Assemblée nationale, vous avez exprimé une préoccupation pour le sort des populations civiles à Gaza, mais l'heure est venue de taper du poing sur la table, car la voix de la France compte encore au Proche-Orient. M. Macron doit prendre la parole fortement en faveur de la paix, comme d'autres l'ont fait par le passé. Vous avez annoncé hier l'ouverture d'un couloir humanitaire : où en sommes-nous ? L'Union européenne, réunie hier soir, est encore divisée, ne bouge pas, ou tergiverse. La violation massive des droits de l'homme et la suspicion de crimes de guerre à sa porte doivent la faire réagir. Beaucoup renvoient dos à dos agresseurs et agressés. Pourtant, les faits, les images, les chiffres démontrent le choix de la guerre et de la violence fait par Benyamin Netanyahou et l'extrême droite israélienne. Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé hier la nécessité d'une solution politique. Allez jusqu'au bout Au-delà d'un hypothétique vote à l'ONU d'un cessez-le-feu sur l'initiative de la France, qui peut s'avérer bien tardif, à moyen et long termes, seule la coexistence pacifique de deux États, israélien et palestinien, ouvrira la voie d'une solution heureuse au Proche-Orient. c'est de tout faire pour la cessation des hostilités et le respect de la souveraineté de Jérusalem-Est en stoppant la politique de colonisation. Il faut absolument faire entendre raison au gouvernement israélien. Monsieur le Premier ministre, quand la France va-t-elle reconnaître l'État palestinien ? Car cette reconnaissance est la clé de la paix

à l'Assemblée nationale, la situation au Proche-Orient est effectivement extrêmement grave et préoccupante. Elle est, vous le savez toutes et tous, la conséquence d'une absence de perspective politique qui n'a que trop duré, et qui continuera à produire de la violence si la volonté n'est pas là pour avancer résolument vers l'établissement de deux États dans le cadre du droit international, des résolutions du Conseil de sécurité et des paramètres agréés.

des familles entières, palestiniennes et israéliennes, endeuillées ; des images de destruction terribles ; une population israélienne qui vit sous la menace des roquettes. Rien de tout cela ne peut nous laisser indifférents. Je veux, comme hier, redire ici l'attachement indéfectible de la France à la sécurité d'Israël. Le Hamas a cherché à récupérer, à instrumentaliser une situation de tension à Jérusalem, au prix de souffrances insupportables pour les populations civiles. La France condamne donc une nouvelle fois par ma voix, avec la plus grande fermeté, les tirs de roquettes par le Hamas et d'autres groupes terroristes depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. Ils sont inacceptables et, le Président de la République l'a rappelé, ils doivent cesser immédiatement. Dans leur réponse militaire, les autorités israéliennes doivent agir de façon proportionnée et dans le strict respect du droit international. Nous sommes inquiets de la situation humanitaire des populations civiles à Gaza, auxquelles l'aide doit parvenir rapidement et sans entrave. Des premières mesures ont été prises en ce sens, et nous agissons, madame la présidente Assassi, puisque telle était votre question, pour qu'elles se concrétisent très rapidement et qu'elles puissent s'amplifier. Enfin, comme je le précisais également hier aux députés, la sécurité du personnel humanitaire et médical, d'une part, et des journalistes, d'autre part, doit absolument être préservée. Le cycle de violence en cours, malheureusement, ne se limite pas à Gaza. Dans plusieurs villes, des heurts entre communautés ont atteint un niveau inédit. En Cisjordanie et à Jérusalem, les affrontements entre Palestiniens, colons et forces de sécurité israéliennes se multiplient. La France appelle solennellement l'ensemble des acteurs à mettre un terme immédiat à toutes les violences, à toutes les provocations et à toute incitation à la haine pour permettre le retour au calme. À Jérusalem, en particulier, la France a exprimé très tôt sa préoccupation à l'égard des tensions, apparues dès le mois d'avril et qui se sont renforcées tout au long du mois de ramadan. Elle n'a cessé de souligner les risques liés à la poursuite de la politique de colonisation.

Comme vous le savez, le Président de la République s'est entretenu au cours des derniers jours avec le Premier ministre Netanyahou et le Président Abbas. Il a rencontré le Président Sissi, dont nous soutenons pleinement les efforts de médiation. réuni hier en visioconférence avec le roi de Jordanie et le même président égyptien pour organiser la convergence de nos efforts. Il s'agit de permettre un accès humanitaire complet à Gaza, la mise en place rapide d'un cessez-le-feu effectif et l'adoption à cet effet d'une résolution du Conseil de sécurité. Ne doutez pas, madame la présidente Assassi, mesdames, messieurs les sénateurs, de la ferme volonté de la France de peser de tout son poids dans cette région du monde, où se déroulent des événements extrêmement graves.

alors que la plupart des États européens poursuivent l'allégement progressif de leurs mesures de restriction, la résurgence de l'épidémie dans plusieurs pays à travers le monde demeure alarmante. Je pense notamment à l'Inde, au Népal ou encore au Brésil. Les épidémies ne connaissent pas de frontières, et la covid-19 ne fait évidemment pas exception. Seule une vaccination rapide, efficace et accessible à tous permettra de surmonter cette pandémie. Pour y arriver, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Alliance Gavi et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies ont lancé l'initiative Covax, un mécanisme mondial devant accélérer la fabrication de vaccins et garantir sa distribution équitable à travers le monde. Grâce à ce dispositif, 64 millions de vaccins ont pu être distribués dans 124 pays. Pourtant, ce lundi, l'Unicef a tiré la sonnette d'alarme sur le retard pris par Covax, estimant que, si les pays du G7 et les États membres de l'Union européenne partageaient 20 % de leurs stocks de juin, juillet et août, alors, plus de 150 millions de doses pourraient être données. Cela sauverait bien des vies dans ces pays en difficulté. La France a été le premier pays à donner 100 000 doses Covax. Quelques semaines plus tard, le Président de la République a appelé les pays anglo-saxons, et au premier rang les États-Unis, à contribuer davantage à la circulation de ces vaccins. Monsieur le secrétaire d'État, puisque le temps joue contre nous, comment accélérer l'initiative Covax et répondre à ce message de solidarité et d'urgence formulé par l'Unicef ? Quel rôle pourrait-on imaginer pour le laboratoire français Sanofi, qui vient de publier des résultats prometteurs ? La parole

vous soulignez l'importance de la solidarité internationale pour lutter contre cette pandémie. Vous avez raison. C'est non seulement notre devoir humanitaire et moral de soutenir les pays, très nombreux aujourd'hui, qui n'ont pas accès, faute de moyens financiers ou de capacités de production, aux vaccins, mais c'est aussi notre intérêt sanitaire, français et européen. En effet, nous voyons bien, devant la prolifération de certains variants, que nous ne serons pas en sécurité tant que le monde entier ne sera pas progressivement vacciné. Nous devons donc accélérer.

Nous devons pour cela mobiliser l'ensemble des vaccins disponibles. Vous évoquiez celui de Sanofi. Le laboratoire a annoncé des résultats positifs en tout début de semaine. Nous espérons, sous réserve que la phase III se déroule bien, que l'autorisation de mise sur le marché puisse être donnée et que ce vaccin complémentaire soit disponible au dernier trimestre de cette année. Cela sera nécessaire pour l'Union européenne, pour la France, car nous en aurons encore besoin, et pour accélérer nos efforts internationaux. Je rappelle aussi que, dans ce souci de solidarité, l'Union européenne a commandé, au total, plus de 2,5 milliards de doses. C'est évidemment beaucoup plus qu'il n'en faut pour vacciner notre propre population, ce qui est bien sûr notre priorité, mais cela permet aussi de donner un certain nombre de doses le plus vite possible. Enfin,

Monsieur le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, malheureusement, une fois encore, l'actualité se fait terrible et terrifiante au Proche-Orient. Les images montrent toutes les misères de la guerre, frappant une population israélienne et palestinienne soumise à la terreur des bombardements et des tirs de roquettes. Ces affrontements sont les plus violents depuis 2014, avec un bilan déjà trop lourd, tant dans la bande de Gaza, qui atteint désormais près de 230 morts, dont 58 enfants, qu'en Israël, qui a recensé 12 victimes, dont 2 enfants, sans compter les blessés dans les deux camps. Le constat est terrible. Alors que les hostilités sont entrées dans leur deuxième semaine, sans aucun signe d'apaisement, puisque les violences s'étendent maintenant à la Cisjordanie, les grands pays occidentaux, mais aussi la Russie, la Chine ou le monde arabe semblent impuissants, à ce stade, à enrayer cette mécanique. Cela pose la question de leur engagement réel, et, partant, du nôtre, monsieur le secrétaire Le secrétaire général de l'ONU a appelé à l'arrêt immédiat des combats, qui risquent de « déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable dans la région ». Les 15 membres du Conseil de sécurité ont condamné les violences contre les civils, des deux côtés, et la presse à Gaza,

Monsieur le secrétaire d'État, n'est-il pas urgent d'agir au nom de la seule raison qui vaille, celle de la paix et de la protection des populations civiles, que la France défend à travers la solution à deux États ? Au-delà de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU, la France est l'un des rares pays à avoir la capacité de parler aux deux parties. Pourtant, elle choisit de soutenir une médiation menée par l'Égypte. N'y a-t-il donc aujourd'hui ni plan de paix ni interlocuteur capable d'en proposer un ? Que penser de la prise de position minimaliste des Européens sur une solution politique, qui n'a même pas fait l'unanimité, et qui nous marginalise tous dans un rôle de soutiens humanitaires, économiques, à défaut d'être des acteurs d'un véritable processus de paix ?

Le Premier ministre a évoqué à l'instant la position d'équilibre que la France défend depuis plusieurs jours de manière active. Vous l'avez dit aussi, nous sommes un des rares pays qui puisse parler aux

car je crois que nous devons aller ensemble dans ce sens. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et nous avons, à ce titre, un rôle clé à jouer pour relayer les efforts de médiation et de désescalade. C'est ce qu'en ce moment même Jean-Yves Le Drian est en train de faire avec une nouvelle réunion du Conseil de sécurité. Comme vous l'avez indiqué, nous avons proposé un projet de résolution, qui vise à amplifier ces efforts diplomatiques et à tenir cet équilibre entre la nécessité d'un accès humanitaire rapide,

ces dernières heures. En effet, quelques partenaires européens n'ont pas voulu jouer ce jeu collectif. Néanmoins, le haut représentant Josep Borrell a été très clair sur le fait que la position européenne était la même que celle que défend la France, c'est-à-dire le soutien à la sécurité d'Israël, l'appel à la désescalade et l'appui à tous les efforts humanitaires d'urgence. Nous poursuivrons ce travail ces prochaines heures avec nos partenaires de la région. Je le répète, nous sommes un des rares pays à pouvoir parler à tous les acteurs régionaux, Jordanie et Égypte en particulier, pour assurer le plus vite possible le retour à un dialogue, le cessez-le-feu et le soutien humanitaire.

L'aménagement numérique est devenu un enjeu majeur de développement territorial dans les zones les plus rurales de notre pays. Le numérique ne cesse d'envahir notre quotidien et cette tendance a été accélérée par la crise sanitaire, qui a accentué son usage sur le plan économique, dans l'accès à l'éducation, aux soins, au travail, aux services publics et aux droits élémentaires. D'après les prévisions de l'Observatoire du très haut débit, 87 % des Français seraient raccordables à la fibre en 2022, alors que l'objectif fixé par le Gouvernement à cette échéance est 80 %. Ces chiffres encourageants reflètent cependant des réalités contrastées. Les zones très denses sont couvertes en très haut débit à hauteur de 85 %, alors qu'au sein des zones de réseaux d'initiative publique, situées en milieu rural, ce taux n'atteint que 32 %. De plus, l'Observatoire estime à plus de 2 millions le nombre de locaux en difficulté pour un raccordement à la fibre dans les zones les plus reculées, où le déploiement est plus long et plus coûteux. Les opérateurs expliquent la lenteur du déploiement par des arguments qui laissent dubitatifs : un manque de techniciens télécoms, malgré des recrutements qui ont dépassé les espoirs de la filière ; un procédé d'adressage encore insuffisant, alors que les communes rattrapent leur retard, avec plus de 3 millions d'adresses créées ; ou encore une réglementation limitant la pose de la fibre du fait de la charge pouvant être supportée par les poteaux pour les lignes aériennes. Par ailleurs, l'accélération du déploiement de la fibre ne doit pas se faire au détriment de la qualité : entre un quart et un cinquième des raccordements finaux se soldent par un échec, les travaux et le matériel étant trop souvent à l'origine de malfaçons ou l'objet de dégradations. ministre, pouvez-vous nous dire quelles actions le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre pour accélérer un déploiement d'un très haut débit de qualité en milieu rural ?

Je vous confirme que le déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné au travers du « New Deal mobile » est bien une priorité du Gouvernement, particulièrement de Cédric O et de mon ministère. Nous avons d'ailleurs déployé depuis le début de ce quinquennat des moyens sans précédent pour accélérer cette transition. Le plan France Très haut débit a ainsi connu une formidable accélération, le pourcentage de locaux raccordables passant de 24 % en 2017

conçu, en dehors des agglomérations, à l'échelle de l'ex-région Auvergne. Entre décembre 2017 et décembre 2020, le pourcentage de logements ou de locaux professionnels raccordables au réseau de la fibre y est, certes, passé de 22 % à 53 %.

afin d'éviter les dégradations. Nous savons qu'il existe aussi des problèmes d'adressage et des difficultés de raccordement complexes à résoudre. Avec l'Arcep et la commission où siège votre collègue sénateur que j'aperçois, nous surveillons tout cela de très près.

lundi 10 mai, le Sénat modifiait le projet de loi constitutionnelle tendant à inscrire à l'article 1 de notre loi fondamentale la garantie de la préservation de l'environnement et de la biodiversité, et la lutte contre le dérèglement climatique. Nous regrettons vivement ce choix de la majorité sénatoriale, qui n'a toujours pas pris la mesure de l'urgence environnementale. En choisissant de s'opposer à la décision souveraine du peuple, elle a confirmé que le gaullisme n'était plus qu'un lointain souvenir. En choisissant de laisser la maison brûler, elle a montré que l'héritage de Jacques Chirac l'était également. Mes chers collègues, à force de regarder ailleurs, vous ne voyez même plus l'évidence. Le choix que vous souhaitez laisser aux Françaises et aux Français n'en est pas un. La rédaction que vous proposez est symbolique, sans portée normative. Un référendum cosmétique n'intéresse personne. De toute façon, maintenant, le calendrier devient intenable : il sera impossible d'organiser un référendum digne de ce nom avant l'élection présidentielle. À en croire les indiscrétions, la veille de notre débat,

sont des impératifs désormais majeurs. Je me faisais la réflexion que, depuis que je suis Premier ministre,

ce référendum pour reverdir le bilan écologique du quinquennat, c'est raté : nous n'en aurons même pas le symbole ! Il s'agit encore d'une promesse présidentielle qui risque de ne pas être tenue, d'une proposition de la Convention citoyenne qui risque d'être mise au panier.

chers collègues, nous y voilà ! Après quinze mois de crise sanitaire et trois confinements, nous voyons enfin le bout du tunnel. L'assouplissement des contraintes sanitaires nous envoie des signes tangibles recul du couvre-feu à vingt et une heures, réouverture des terrasses, des musées, des cinémas et de tous les commerces. J'ai bon espoir que les Français se ruent dès aujourd'hui dans les petits commerces, car ils ont reporté bon nombre de leurs achats. Les commerçants, eux, ont besoin de renouer le contact avec leurs clients pour écouler leurs stocks et reconstituer leurs marges. Je l'ai dit : les Français attendaient ce jour depuis longtemps, et on les comprend : ils vont pouvoir, de façon très progressive, retrouver tout ce qui fait le sel de la vie. Nous partageons tous cet engouement. Mais ce retour progressif à la normale ne doit pas conduire à confondre vitesse et précipitation. C'est ce que souhaitent les commerçants qui nous ont sollicités, et je tiens à associer à ma question ma collègue Vanina Paoli-Gagin. Les commerçants vont reprendre leur activité et se réhabituer à travailler Il faut que les recettes commerciales remplacent peu à peu les aides publiques. C'est dans ce contexte que se pose la question des soldes d'été, qui doivent débuter le 23 juin. De l'avis des petits commerçants- j'ai encore parlé ce

Les policiers nous protègent, mais l'État n'est plus capable de les protéger. Ils ont peur. Leur émotion, leur indignation, leur colère se sont exprimées dans la dignité il y a tout juste deux heures.

mais les mots ne suffisent plus : il faut que vous changiez de logiciel ! On l'a fait ! Il faut instaurer des peines minimales automatiques contre tous les agresseurs des forces de l'ordre et de sécurité. Monsieur le Premier ministre, allez-vous réellement assurer la protection et la sécurité des policiers en décrétant l'urgence de la réponse pénale

dans l'enceinte même de l'établissement. Je souhaiterais conclure en disant que la réalité du travail des policiers et des gendarmes n'est souvent pas celle qui est décrite dans les médias et sur les plateaux de télévision. À 400 reprises, chaque semaine, des policiers et des gendarmes interviennent pour sauver la vie de femmes et d'enfants confrontés à des violences intrafamiliales. Mais ce n'est pas la

Christian Cambon, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, les plaies du conflit meurtrier au Haut-Karabagh sont encore ouvertes que l'Azerbaïdjan multiplie les provocations contre l'Arménie refus honteux de libérer les prisonniers de guerre, destruction méthodique du patrimoine culturel et religieux des territoires arméniens qu'il contrôle. La situation s'aggrave encore avec l'incursion de 350 soldats azéris, qui se sont carrément installés sur le territoire arménien autour du lac Noir et de la zone de Verin Shorzha.

l'attaque du Haut-Karabagh était la première étape d'un plan de l'Azerbaïdjan et de la Turquie visant à établir une continuité territoriale entre eux aux dépens de l'intégrité de l'Arménie. Le Président de la République a immédiatement appelé au retrait des troupes

le groupe de Minsk dont la France assure la coprésidence ? Allez-vous saisir le Conseil de sécurité de l'ONU ? Il s'agit de défendre nos valeurs et notre amitié de toujours avec le peuple arménien. En d'autres termes, face à ce drame, allez-vous passer de la diplomatie des déclarations à la diplomatie de l'action ?

il y a eu ces derniers jours une nouvelle montée des tensions et, vous l'avez rappelé, l'incursion extrêmement préoccupante de troupes azerbaïdjanaises dans une région arménienne, celle du Syunik. Des troupes ont pris position dans une zone où la frontière internationale est mal définie et se sont introduites sur le territoire arménien. Cet incident montre que le cessez-le-feu reste extrêmement fragile et que nous ne pourrons pas faire l'impasse sur un règlement global du conflit. La France y prend sa part dans le cadre du groupe de Minsk, dont nous assurons, vous l'avez rappelé, la coprésidence. C'est dans ce cadre privilégié que nous poursuivrons nos efforts pour aboutir au règlement politique du conflit. La libération de quelques prisonniers arméniens par l'Azerbaïdjan était un pas important dans le sens de l'apaisement, mais c'est aujourd'hui sans nul doute à l'Azerbaïdjan qu'il appartient d'aller plus loin et de montrer des signes concrets de désescalade. Nous sommes mobilisés à tous les niveaux pour assurer ces efforts diplomatiques. Le Président de la République s'est entretenu avec le Premier ministre arménien le 13 mai. Jean-Yves Le Drian s'est entretenu avec ses homologues d'Arménie et d'Azerbaïdjan ces derniers jours, avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, pour

Madame la ministre, le 3 septembre dernier était présenté le plan de relance de 100 milliards d'euros dont la territorialisation devait être un gage d'efficacité, d'adaptabilité, d'équité et de cohésion. Sur le total, 10,5 milliards d'euros doivent profiter aux collectivités locales. Un premier bilan indique que 5,3 milliards d'euros ont déjà été mobilisés, mais il fait également apparaître de grandes disparités entre les territoires. Ainsi, alors que la moitié de l'enveloppe a été distribuée, certains départements ne bénéficient

disposent de l'arsenal administratif nécessaire pour traiter rapidement les dossiers. En revanche, les plus petites collectivités, qui ont pourtant été un maillon important dans la gestion de la crise sanitaire, rencontrent des difficultés pour monter les dossiers faute d'ingénierie, de technicité et d'un accompagnement suffisant. Ensuite, le dispositif est trop complexe : les programmes développés sont multiples et marqués par des critères qui deviennent vite restrictifs. Ils traduisent une absence de souplesse, dont les élus de terrain ont désespérément besoin. Quant aux départements, en particulier les plus petits, soumis aux contrats de Cahors et à de fortes contraintes financières et qui ont en conséquence des programmes d'investissement limités, ils n'ont pas été en mesure de présenter au pied levé des projets chiffrés dont les travaux doivent être achevés en 2022. Cette situation ne peut perdurer sans créer inévitablement un plan de relance à deux vitesses. La fracture entre nos territoires les plus pauvres, notamment ruraux, et nos territoires les plus riches est déjà assez grande sans que le plan de relance vienne l'exacerber.

Cette année, les candidats ont donc postulé Parcoursup et ont dû joindre des « écrits personnels » à leur candidature. Les centres d'intérêt et l'opinion personnelle des candidats semblent désormais devenus aussi importants que la maîtrise des savoirs académiques, que le concours anonyme permettait de vérifier de manière objective.

recrutement permet à tous les jeunes de notre pays qui en ont les capacités de rejoindre cette école. C'est le principe même de la sélection. Les nouvelles règles d'admission à Sciences Po se déclinent autour de quatre blocs.

Madame la ministre, j'aurais tellement voulu que vous répondiez à ma question ! Depuis la création de Polytechnique, la République a choisi des concours pour départager les meilleurs. Anonymes, organisés pour tous et dans les mêmes conditions, les concours sont l'essence de la méritocratie républicaine. Pourtant, les voilà contestés : ils pénaliseraient les candidats qui ne sont pas assez scolaires ! Cette petite musique bien-pensante fait dire à Pascal Perrineau que « Sciences Po est en proie à une fascination américano-centrée oublieuse de l'histoire intellectuelle de la maison ». Pour répondre à cette pensée militante, les candidats devront-ils se conformer aux lubies d'une direction plus obnubilée par son image et plus soucieuse de singer un pseudo-modèle américain que de former les élites de la Nation ? Plus généralement, devront-ils chercher à s'épanouir dans les engagements à la mode pour répondre aux canons d'éphémères pensées dominantes ? Bref, le fait d'être un

car ils subissent en outre les nombreux dysfonctionnements de la réforme de l'accès aux études de santé. Soyons clairs : les objectifs initiaux de la réforme sont les bons. Alors que la Paces conduisait à une catastrophe pédagogique et humaine, la réforme a été construite.

comme en témoignent les nombreuses auditions des parties prenantes dans le cadre de la mission d'information dont j'ai été rapporteure, cette réforme complexe a été trop vite appliquée, insuffisamment préparée et pilotée. Il n'y a eu, pour ces milliers d'étudiants, ni lisibilité, ni transparence, ni équité. J'espère que les correctifs nécessaires seront apportés à l'avenir. Je souhaite évoquer plus particulièrement la situation de la promotion actuelle. Celle-ci a « essuyé les plâtres » et se trouve dans une situation très difficile sur les plans universitaire, psychologique et humain. étudiants attendaient légitimement clarté, justice et bienveillance, on leur a répondu à coups de chiffres et de quotas ... Et si tard ! Pour eux, il est évident que l'objectif initial de réussite n'a pas été atteint.

les chiffres que vous annoncez sont répétés comme des mantras depuis le début. Pour ma part, je vous parle du terrain, des milliers d'étudiants et de l'urgence. Où est la réussite

Je voudrais évoquer un temps que les moins de 4 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où votre majorité défendait avec force l'interdiction du cumul des mandats ; un temps où les « marcheurs » voulaient incarner la rupture avec l'ancien monde, c'est-à-dire avec les pratiques politiques qu'ils jugeaient d'un autre temps.

La parole est à M. le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne.

Premier ministre. Après de nombreux débats, je me félicite que, jour après jour, les ralliements à l'instauration d'un minimum jeunesse ou d'un revenu d'urgence pour les jeunes se multiplient. Alors qu'au début de l'année je n'ai essuyé que des refus, j'observe, aujourd'hui, que beaucoup de formations politiques trouvent légitime cette proposition, même dans les rangs de la majorité gouvernementale. Je fais référence bien évidemment à M. Laurent Saint-Martin, tête de liste de La République En Marche en Île-de-France, qui propose un dispositif similaire. Autrement dit, la question n'est plus de savoir si nous devons le faire, mais comment vous allez procéder pour le mettre en oeuvre

Ce n'est pas moi qui le dis, mais le haut-commissaire au plan, M. Bayrou, dans son récent rapport. Il manquerait 40 000 à 50 000 naissances par an pour assurer le renouvellement de nos générations.

En décembre 2020, un médicament innovant, le Trodelvy, est devenu accessible en France pour les femmes atteintes d'un cancer du sein « triple négatif » métastatique. Ce médicament a obtenu une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) nominative : c'était une excellente nouvelle pour les patientes.

sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Compte tenu

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (projet n° 535, texte

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, notre droit national s'enrichit régulièrement de dispositions décidées conjointement avec les autres États membres de l'Union européenne. Créer un cadre unifié sur de nombreux sujets en Europe

C'est tout l'enjeu du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances

Certaines mesures sont de portée générale et dans la continuité des règlements passés, d'autres permettent de sanctuariser de réelles avancées, certaines d'entre elles étant défendues depuis 2017 par le Gouvernement et sa majorité. Permettez-moi ainsi de m'arrêter plus spécifiquement sur ces dernières.

Ainsi, le renforcement du cadre social pour le transport routier est l'une des avancées majeures de ce texte. Les articles 22 et 23 transposent ainsi l'une des trois parties du paquet mobilité, qui a été adopté l'année dernière par le Parlement européen. Ces mesures sont très attendues, par les transporteurs comme par les élus.

sur le sujet. Je pense aussi à l'amélioration des conditions de travail des conducteurs, avec de nouvelles sanctions pour les entreprises qui ne respecteraient pas le droit au retour des conducteurs dans le pays d'établissement ou à leur domicile et le durcissement des sanctions en cas de non-respect des conditions de repos. encore au renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale dans le transport routier de marchandises pour limiter le cabotage systématique par les transporteurs étrangers. Il sera en effet nécessaire de respecter une période de carence de quatre jours entre deux périodes de cabotage. Le secteur maritime est aussi concerné- c'est l'objet des articles 16 à 21 -, avec des évolutions dans la formation, le temps de travail et la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à pension des marins. Cette mesure est par exemple essentielle à la signature d'accords relatifs à l'activité partielle de longue durée (APLD) dans le secteur. Ce texte permettra également plusieurs avancées techniques et innovantes pour les transports. C'est l'enjeu de la refondation de la réglementation sur le service européen de télépéage. Ce dispositif doit permettre de fluidifier le trafic, d'améliorer l'interopérabilité technique des dispositifs de télépéage européens et de renforcer la lutte contre la fraude en facilitant l'échange transfrontalier d'informations sur les véhicules et les propriétaires fraudeurs. L'Europe et la France doivent aussi être à la pointe de l'innovation. C'est l'objectif d'une meilleure régulation de la teneur en soufre dans les combustibles marins à l'article 16, essentielle pour la transition écologique du secteur. C'est aussi la visée d'un développement contrôlé des activités aériennes, avec l'introduction d'un régime de déclaration, concernant concernant notamment les opérations de drones. Je mentionne également quelques enjeux territoriaux, en particulier liés au secteur aérien et au Brexit, qui seront réglés grâce à ce texte.

Je sais que le Sénat y est attaché et cela a fait l'objet de nombreuses questions et amendements que nous évoquerons tout à l'heure. Il s'agira également de prévoir l'extension possible des délégations de service public public pour des lignes aériennes reliant la France à un autre pays européen. C'est l'objet de l'article 7. En matière de sûreté aérienne, un régime approprié de sanctions pénales en cas d'intrusion en zone « côté piste » d'un aérodrome afin d'assurer le respect de la réglementation européenne est aussi proposé à l'article 10. Enfin, le cas particulier de plusieurs aménagements liés au Brexit aux abords du tunnel sous la Manche sera régularisé à l'article 24. Outre les adaptations au droit européen en matière de transport, ce texte comporte également des mesures visant à renforcer la solidité de notre droit environnemental. Sans être exhaustive, je cite l'article 25, qui met en conformité notre régime de sanctions applicables aux violations des règles européennes en matière de mercure. L'article 26 fait de même pour les fluides frigorigènes. L'article 28 présente une importance particulière. Il traduit des mesures relatives au devoir de vigilance des importateurs de métaux et minerais, afin de lutter contre l'importation de substances qui ont financé des conflits armés ou des atteintes aux droits humains. Les articles 29 et 30 toilettent notre droit en matière de droit de l'eau. L'article 31, quant à lui, permet de transposer complètement la directive Habitats pour la partie qui porte sur le suivi des captures et mises à mort accidentelles de certaines espèces protégées. L'article 32, qui est très important à mes yeux, met en adéquation le droit français avec le droit européen pour ce qui concerne l'information environnementale. Enfin, dernière partie, ce projet prévoit des dispositions relatives à la directive Solvabilité II, ainsi que des dispositions relatives au secteur financier et à la protection des consommateurs en matière financière. Ce projet de loi prévoit donc la transposition de dispositions particulièrement importantes sur lesquelles le Gouvernement s'est engagé. Il permet notamment de renforcer notre droit et nos exigences sur des thématiques qui seront au coeur de la prochaine présidence française du Conseil de l'Union européenne, comme le volet social dans le secteur des transports. Sur ces sujets, nous poursuivrons le travail avec le Sénat.

le texte élaboré par la commission sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Compte tenu de la diversité des sujets abordés, trois commissions ont été saisies de ce texte, chacune apportant son expertise et sa complémentarité dans ses domaines de compétence respectifs. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a ainsi examiné trente et un articles, un article ayant été délégué à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et dix articles ayant été confiés à la commission des finances. Les articles examinés par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable portent sur trois domaines : les transports- aérien, routier et maritime -, la prévention des risques et la protection de l'environnement. Dresser un panorama complet du projet de loi qui nous est soumis n'est pas chose facile, tant les sujets abordés sont techniques, spécifiques et nombreux. Dans les interstices de cette complexité, nous avons décelé des sujets de fond aux implications très concrètes pour certains acteurs de terrain, comme les personnels navigants aériens ou les gens de mer, que nous aurons l'occasion d'évoquer plus en détail.

axe -, ce texte vise à préparer la présidence de la France au Conseil de l'Union européenne, qui débutera au premier semestre 2022. Durant six mois, notre pays sera au tout premier plan de la scène européenne. Il s'agit de lui permettre d'assumer ses responsabilités avec cohérence et exemplarité. Il y a bien longtemps, au début des années 2000, notre pays était l'une des lanternes rouges de la transposition du droit européen, avec 176 directives en retard d'intégration.

le Gouvernement et l'administration allaient parfois négocier à Bruxelles des directives, puis semblaient, dans certains cas, se dérober face aux mécontentements qu'ils auraient dû affronter au moment de leur transposition en droit interne. La situation a bien changé, vous l'avez rappelé, madame la secrétaire d'État. La France est désormais parmi les champions d'Europe de la transposition, si vous me permettez cette expression. Je me réjouis de cette évolution, dans laquelle je souhaite que s'inscrive le projet de loi qui nous est soumis. C'est la raison pour laquelle notre commission a souhaité modifier ce texte pour garantir un respect encore plus rigoureux de nos obligations européennes. Ainsi, à l'article 16, qui vise à mieux encadrer la teneur en soufre des combustibles marins, commission a adopté un amendement visant à préciser explicitement que les navires qui fonctionnent en système ouvert et qui rejettent du soufre dans la mer doivent respecter le plafond de teneur en soufre maximale de 3,5 %, comme l'exige la directive européenne. À l'article 20, qui porte sur le travail des jeunes à bord des navires, la commission a comblé une importante lacune de transposition. Le droit européen prévoit en effet que ces jeunes ont droit à un temps de pause quotidien. Le droit français prévoyait cette garantie, qui a été abrogée par erreur, par voie d'ordonnance, en 2010. À l'unanimité, la commission a décidé de réintroduire ce temps de pause dans notre droit. Cet exemple démontre, une fois de plus, que le recours aux ordonnances s'accompagne bien souvent d'une moindre qualité normative. Le constat est d'autant plus alarmant que l'article 20 vise aussi à revenir sur une ordonnance ayant modifié, au mois de septembre dernier, le cadre juridique de la période de travail de nuit à bord des navires d'une manière non conforme à la directive européenne. Or on ne peut laisser subsister instabilité et incertitudes juridiques ni contourner le Parlement dans un domaine aussi sensible que les conditions de travail de mineurs. une fois de plus, mes chers collègues, pour un examen vigilant des demandes d'habilitation qui nous sont adressées par le Gouvernement. Ensuite- et c'est le deuxième axe -, plusieurs articles visent à atténuer les effets de la crise sanitaire et du Brexit. J'en citerai deux. l'article 19 a pour objet de permettre le maintien de la possibilité pour les ferries qui naviguent entre la France et le Royaume-Uni d'exploiter des casinos en dépit du Brexit. Depuis la loi pour l'économie bleue de 2016, il est possible d'exploiter des casinos flottants sur les lignes intracommunautaires. Cette mesure, introduite par un amendement adopté dans cet hémicycle, visait à renforcer la compétitivité de la flotte française face à la concurrence étrangère, notamment britannique. Les machines à sous sont essentielles à l'équilibre financier des compagnies de ferries françaises, actuellement frappées de plein fouet par la crise et le Brexit. Je vous propose le maintien de cette mesure qui s'inscrit dans la continuité de la position qui était la nôtre lors de son introduction en 2016. part, l'article 21 concerne l'impact de la crise sanitaire pour les marins. Depuis le mois de mars 2020, près de 8 000 marins ont été placés en activité partielle dans notre pays. Cet article soumet les périodes d'activité partielle effectuées par des marins au versement de cotisations vieillesse, afin d'atténuer les effets de la crise sur le montant de leur retraite. C'est une avancée sociale que je tiens à saluer.

Au cours des auditions, des gens de mer m'ont fait part de la situation de certains de leurs collègues qui devront retarder leur départ à la retraite afin que le montant de leur pension ne soit pas affecté. Cette situation me préoccupe et j'aurais déposé un amendement sur ce point si l'article 40 de la Constitution me l'avait permis. Il n'est pas souhaitable que certains marins, déjà fortement éprouvés par le contexte actuel, se retrouvent à devoir travailler plus longtemps pour compenser les effets de la crise, situation qu'ils n'ont pas choisie. D'après les informations que j'ai pu recueillir, quelques dizaines de personnes tout au plus seraient concernées.

Comme je vous l'ai indiqué, notre commission a gardé à l'esprit le contexte de crise tout au long de ses travaux, en veillant à protéger plus efficacement certains acteurs particulièrement fragilisés. Ainsi, s'agissant du volet aérien du projet de loi, les personnels dont nous avons rencontré les représentants s'inquiètent des conditions de mise en oeuvre du nouveau dispositif de tests, portant non pas sur l'alcool ou les stupéfiants, mais sur des substances psychoactives parfois prescrites par un médecin. du secret médical et de la vie privée ? également des « faux positifs » dont la pandémie a rappelé l'existence ? Nous proposons d'approuver l'habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce sujet compte tenu des garanties offertes par le dispositif, mais nous soulignons la nécessité de respecter le secret médical et d'agir avec tact, surtout et y compris dans la période dramatique que traverse aujourd'hui le secteur aérien. les personnels navigants sont rassurés par le renforcement des sanctions prévues pour les passagers indisciplinés, dits PAXI dans la langue des conventions internationales. Le décuplement des incidents en vingt ans relevé dans les statistiques correspond malheureusement à une réalité de terrain ; les incivilités et les violences doivent cesser. Enfin- et c'est le troisième axe de nos travaux je vois dans ce texte un prélude aux débats que nous aurons dans les prochaines semaines lors de l'examen du projet de loi Climat et résilience. En effet, il comprend sept articles relatifs à l'environnement et à la prévention des risques. J'en citerai deux. L'article 26 vise à garantir le respect du système de quotas conçu par l'Union européenne pour réduire la circulation de fluides frigorigènes, ces substances que nous retrouvons quotidiennement dans nos réfrigérateurs ou systèmes de climatisation et qui ont un pouvoir de réchauffement climatique entre 1 000 et 15 000 fois plus puissant que le CO2. À l'article 16, que j'ai déjà cité, qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins, nous avons adopté un amendement visant à préciser que les méthodes mises en oeuvre sur certains navires afin de réduire les émissions de soufre ne peuvent avoir d'incidence négative sur l'environnement. Notre objectif est de lutter plus efficacement contre les, ces systèmes d'épuration qui permettent à certains navires de filtrer les polluants au niveau des cheminées afin de respecter les normes de pollution de l'air, pour ensuite les rejeter à la mer. Ces sont un véritable fléau pour les écosystèmes marins. Selon l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ils seraient responsables de 78 % des rejets en mer. Telles sont les trois logiques qui ont irrigué nos travaux : assurer l'exemplarité de la France sur la scène européenne, atténuer les effets de la crise, renforcer la protection de l'environnement. J'ajouterai un dernier point : notre commission a souhaité garantir une meilleure transparence économique du secteur aéroportuaire. Elle a donc adopté un amendement permettant de conforter les pouvoirs de l'Autorité de régulation des transports, en prévoyant un pouvoir de collecte des informations dans le domaine aérien analogue à ce qui existe pour le transport ferroviaire. Mes chers collègues, avant de conclure, je souhaite mentionner le groupe de travail sur la modernisation des méthodes de travail du Sénat, qui a récemment rendu ses conclusions. Le groupe de travail a dressé le constat de la hausse massive du recours aux ordonnances et appelé à une réappropriation, par le Parlement, de ses prérogatives en matière de ratification. Notre commission a ainsi voulu saisir l'occasion offerte par ce texte pour montrer l'exemple, en introduisant un article 24 proposant la ratification de six ordonnances prises sur le fondement de la LOM en 2020 et 2021. La parole

la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a bien voulu déléguer à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées l'examen sur le fond de l'article 28 relatif aux minerais de conflit. Je l'en remercie, car le règlement européen qui nous est soumis vise à adapter en droit national le contrôle du devoir de diligence des importateurs de l'Union européenne à l'égard de la chaîne d'approvisionnement de l'étain, du tantale, du tungstène et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. C'est un sujet qui concerne notre diplomatie, mais aussi notre industrie de défense. Tout d'abord, il faut se féliciter de cette étape importante dans la lutte contre le financement des guerres civiles et des groupes armés non étatiques par le commerce de ces minerais. Elle marque l'aboutissement de plus d'une décennie de négociations internationales et européennes. Ce règlement s'inspire de la prise de conscience internationale qui avait conduit, au début des années 2000, les pays de la région des Grands Lacs africains, puis l'Organisation des Nations unies, à lutter contre le trafic des « diamants du sang » et ses conséquences dévastatrices pour les populations. Le règlement européen impose aux importateurs un devoir de diligence pour assurer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et la traçabilité de ces minerais, qui sont indispensables à l'industrie, à l'électronique, aux équipements civils, mais aussi militaires. Il s'agit d'un mécanisme juridique différent de la prohibition ou de l'embargo. Au lieu d'évincer des régions entières du commerce international, au risque d'engendrer davantage de fraudes et de fragiliser encore plus les populations, il place directement les entreprises devant leur responsabilité sociale et leur devoir d'information du client et du public. Le règlement repose donc sur une logique de, c'est-à-dire de conformité au devoir de diligence. Le Gouvernement propose de mettre en place un système de contrôles privilégiant l'incitation par rapport à la sanction. En cas de manquement, l'autorité administrative pourra enjoindre aux intéressés d'appliquer des mesures correctives sous peine d'exécution d'office et d'astreintes administratives pouvant aller jusqu'à 1 500 euros par jour de retard. On peut s'interroger sur l'efficacité d'un tel dispositif dépourvu de sanction pénale, mais nous avons considéré qu'il n'y avait pas lieu sur ce point de « suradapter » notre législation. Par ailleurs, il faut reconnaître deux vertus à ce règlement. Sa première vertu est de contrôler le commerce de ces quatre minerais. C'est un dispositif européen porteur d'espoir, qui ouvre aussi une réflexion, sous un angle environnemental, concernant d'autres secteurs, dans le domaine des terres rares et de minerais comme le cobalt, nécessaire à la fabrication des batteries. La seconde vertu, qu'il faut signaler, est la clause de « revoyure » prévue en janvier 2023 pour que la Commission européenne réexamine l'efficacité du dispositif et étudie la nécessité ou non d'adopter des mesures plus contraignantes. Pour conclure, je vous propose d'adopter l'article 28 du présent projet de loi tel que nous l'avons modifié en commission, d'une part pour préciser le périmètre des contrôles sur la documentation devant être tenue par les importateurs, d'autre part pour nous assurer de la proportionnalité du montant des astreintes administratives à la gravité des manquements et à la situation financière des entreprises. La parole

sans doute pour démontrer son exemplarité en matière de transposition, alors que la France s'apprête à prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne au début de l'année prochaine, le Gouvernement a décidé de recourir à un « texte balai » d'adaptation au droit de l'Union européenne. Si l'on peut parfaitement comprendre cette volonté, il en résulte inévitablement un texte touffu et technique portant sur de nombreux domaines. La commission des finances dispose sur ce texte d'une délégation au fond pour le dernier des cinq chapitres, qui rassemble les dix articles portant sur le droit économique et financier. On peut distinguer, parmi ces articles, deux catégories. La première comporte des dispositions techniques visant à remédier à des difficultés d'explication et d'articulation avec les règles européennes existantes. Celles-ci font donc suite à de précédentes transpositions en droit interne ou à des aménagements décidés pour préparer le Brexit. C'est le cas des articles 33, 37, 38, 39, 40 et 42. Ces articles, de nature essentiellement technique, ne nous ont pas paru poser de difficultés. La commission des finances a donc adopté uniquement trois amendements rédactionnels et de coordination. La seconde catégorie d'articles rassemble, à l'inverse, des dispositions visant à adapter notre droit économique et financier à de nouvelles évolutions du droit de l'Union européenne. C'est le cas des articles 34, 35, 36 et 41. Sur les quatre articles, deux procèdent à des transpositions « en dur », tandis que deux autres sollicitent une habilitation à recourir aux ordonnances. Ainsi, les articles 34 et 35 transposent directement deux articles d'une même directive de 2019 qui mettent en oeuvre les conclusions de l'exercice de revue des autorités européennes de supervision mené en 2019. Ils ne soulèvent pas de difficultés et ont seulement fait l'objet d'amendements rédactionnels en commission. En ce qui concerne les deux articles sollicitant une habilitation à légiférer par ordonnance, nous avons fait preuve d'une grande vigilance, en vérifiant qu'ils se justifiaient par l'absence de marge de manoeuvre du législateur et l'impossibilité d'intégrer directement dans la loi les mesures de transposition. Il nous a semblé que ces deux conditions étaient pleinement remplies pour l'article 36, qui vise à transposer la série de mesures de relance par les marchés de capitaux contenues dans la directive 2021/338 du 16 février 2021. À l'inverse, l'article 41 nous a paru emporter un risque majeur de dessaisissement du Parlement. Il visait en effet initialement à habiliter le Gouvernement non seulement à mettre notre droit national en conformité avec le nouveau règlement européen sur le financement participatif, mais également « à adapter et moderniser », notion très large, les dispositions encadrant les activités de financement participatif ne relevant pas du droit européen. En effet, le règlement européen n'encadre qu'une partie des activités de financement participatif aujourd'hui admises en droit interne. Or cette habilitation très large pourrait permettre au Gouvernement de durcir les conditions d'exercice et même de supprimer certaines activités de financement participatif qui n'entrent pas dans le cadre européen. De tels choix très lourds en termes de conséquences pour les acteurs concernés et nullement imposés par le législateur européen doivent faire l'objet d'un débat public et nous semblent relever par essence d'un vote au Parlement. Aussi, pour éviter tout dessaisissement du Parlement, la commission des finances a adopté un premier amendement visant à restreindre le champ de l'habilitation à la mise en conformité avec le règlement européen et à des évolutions ciblées des activités nationales pour l'ouverture des financements participatifs aux sociétés civiles agricoles, mais également pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il s'agit, par cet amendement, de contraindre le Gouvernement à préserver les activités non régulées par le droit européen.

Si les collectivités territoriales peuvent déjà recourir au financement participatif, elles le peuvent uniquement pour financer un service public culturel, éducatif, social ou solidaire. Ce champ nous paraît inutilement restrictif au regard de la variété des projets susceptibles d'être financés. En outre, il existe aujourd'hui une incertitude juridique sur la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir au financement participatif en émettant des obligations. Cet amendement répond donc à une préoccupation exprimée de longue date par les élus, notamment par l'Association des maires de France. Au total, mes chers collègues, la commission des finances a donc adopté sept amendements, dont deux de fond.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, alors que la France s'apprête à prendre la présidence de l'Union européenne,

Quatre ordonnances sont ainsi prévues dans le seul titre premier sur le transport aérien, ce qui semble tout de même beaucoup. Notons ensuite que l'exercice est quelque peu frustrant pour les parlementaires que nous s'agissant le plus souvent de transpositions de règlements européens avec peu de marges de manoeuvre ou de directives techniques, ce qui limite d'autant la capacité d'intervention du Parlement. Je souhaiterais également évoquer l'avis du Conseil d'État, qui déplore « que certaines consultations sont réalisées trop tardivement pour être correctement prises en compte, telle celle de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) requise pour un article du chapitre II, qui s'est réunie le 1 avril et dont l'avis n'a été reçu que le 7 avril, et celle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), qui a été saisie en urgence le 26 mars et devait se prononcer dans un délai de onze jours. Convenons qu'une telle précipitation n'est guère favorable au plein exercice parlementaire. Sur le fond, les mesures de ce projet de loi sont cosmétiques ou sans grandes conséquences. Ainsi, la plupart sont déjà mises en oeuvre en pratique. Par ailleurs, quelques autres mesures nous apparaissent problématiques et les travaux en commission n'ont pas totalement levé nos inquiétudes.

! Pour évoquer encore la question maritime dans sa dimension sociale, nous regrettons que notre amendement à l'article 21 sur la prise en compte de toute la période effective d'activité partielle dans le calcul du droit à la retraite

Enfin, les problématiques du détachement et du cabotage sont évoquées, mais les mesures proposées sont extrêmement faibles pour répondre aux enjeux de rééquilibrage modal et confirment la concurrence assez déloyale de la route, faute là encore de moyens au sein des directions concernées pour faire respecter une réglementation déjà bien faible. Mes chers collègues, pour l'ensemble de ces raisons, et nonobstant le travail assez exhaustif conduit par M. le rapporteur,

Cet accord a été éprouvant pour l'ensemble des parties et demande encore de nombreux ajustements dans des domaines comme le transport ou bien la pêche, pour n'en citer que quelques-uns. Il nous faut aujourd'hui, alors qu'elle traverse une zone de turbulences sans précédent, consolider l'Europe de demain à vingt-sept États membres autour de notre projet commun. Car, outre la perte de l'un de nos membres, la période est plus que singulière : il nous faut faire face à l'épidémie du coronavirus dans laquelle le monde entier se débat encore, plus d'un an et demi après son apparition. Cette crise sanitaire et sociale a eu des conséquences de tous ordres, à commencer par la restriction des libertés, l'un des fondements du projet européen, mais aussi sur nos modes de vie, sur l'État de droit et l'économie. Elle porte atteinte au coeur même de nos ambitions européennes. Cette crise sans précédent a mis en exergue la vulnérabilité de l'Union et ouvre les yeux sur les impératifs de résilience et d'autonomie stratégique. Ainsi, la relance européenne est sans doute une chance unique pour consolider la construction de l'Union, surtout pour sortir plus forts de la pandémie, transformer nos sociétés, créer de nouvelles opportunités et répondre ainsi aux impératifs environnementaux. doit être plus soudée que jamais face aux défis exceptionnels auxquels nous sommes confrontés. L'harmonisation est, me semble-t-il, l'une des clés de voûte de notre performance. Le projet de loi que nous examinons est bien désigné par son titre il agrège un ensemble divers de mesures qui permettra à la France de montrer patte blanche à la veille de sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Sa cohérence ne tient guère qu'à l'adaptation de notre droit aux évolutions législatives décidées par les législateurs européens. Il est hétérogène et technique, mais essentiel pour garantir la bonne application des réglementations européennes. Dans sa version actuelle, je le rappelle, le texte transpose douze directives à travers quarante-deux ont été examinés par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Toutefois, s'il est de coutume que les projets de loi sur les diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne soient complexes, techniques et hétéroclites, ils ne devraient pas être inscrits à l'ordre du jour dans des délais aussi courts, alors que le calendrier est déjà bien chargé. Les conditions d'examen sont discutables, vu l'ampleur et l'importance des sujets traités. Je me contenterai donc de passer rapidement en revue quelques dispositions particulièrement importantes, dont certaines auront des conséquences concrètes. Sur l'aérien, la sécurité et la sûreté seront renforcées, mais il est impératif de voter cette transposition à condition que les pilotes puissent bénéficier non seulement du secret médical, mais aussi de mesures de contre-vérification des tests de dépistage d'alcool ou de psychotropes. Notre groupe a proposé a proposé un amendement en ce sens à l'article 1 du texte. Concernant les télépéages, au regard de l'agitation et de l'effervescence du Gouvernement engagé dans la lutte contre le changement climatique, je trouve paradoxal que notre pays transpose des dispositions européennes contradictoires avec le projet de loi Climat et résilience que nous étudions actuellement. Vous validez, par la transposition de la directive concernant les télépéages, la volonté d'harmoniser un système européen. Cela montre à quel point votre approche régionale régionale de l'écocontribution poids lourds dans le projet de loi Climat et résilience est « micro ». Vous fabriquez un dispositif « puzzle », ingérable tant pour les régions que pour les transporteurs et en contradiction complète avec ce que vous nous proposez de valider dans ce texte. Pour autant, cette directive représente tout de même la première fondation d'une approche européenne, en attendant l'eurovignette poids lourds., la position du Gouvernement n'est pas très claire. Sur le détachement des travailleurs routiers, la transposition des nouvelles règles encadrant le transport routier était très attendue, à la suite des longues négociations relatives au paquet mobilité, qui ont duré plus de trois ans. Cette disposition permettra, je l'espère, d'améliorer concrètement les conditions de travail des chauffeurs routiers, la régulation des règles de cabotage, notamment face à la distorsion de concurrence résultant des réglementations des pays de l'Est, mais aussi du détachement des transporteurs routiers. En juillet dernier, le Parlement européen votait le paquet mobilité pour le transport routier. Malgré les mesures en cours, de nombreuses lacunes et difficultés d'exécution persistaient autour de la législation européenne, avec une application différente entre les États membres. Ce nouveau cadre juridique et le train de mesures sur la mobilité que nous allons valider permettront une meilleure application des règles. Vu la complexité de l'harmonisation et de la clarification des règles sur le détachement des conducteurs, il est nécessaire d'instaurer une application plus ferme des règles spécifiques à ce secteur. secteur. Cette application assurera un équilibre entre, d'une part, la liberté des opérateurs des services transfrontaliers et, d'autre part, de bonnes conditions de travail et de protection sociale pour les conducteurs, dont la nature du travail reste difficile. Cette réforme donnera enfin des conditions sociales décentes aux transporteurs routiers. Effectivement, c'est un sujet politique majeur que le président Emmanuel Macron avait enfourché en début de mandat, allant jusqu'à affirmer qu'il allait tout régler.,

et de sa présidente, Karima Delli, de nombreux progrès ont été portés au paquet mobilité, bien qu'un peu tardivement, ce que je regrette. Les distorsions de concurrence des dernières années ont déjà beaucoup épuisé les transporteurs nationaux. Ce texte présente un progrès sur les conditions de travail et les obligations de retour au pays pour limiter le cabotage, mais aura-t-on des moyens de contrôle suffisants et significatifs ? On attend sur ce sujet une réponse Au sujet du littoral, je tiens à saluer la mise en place d'exemptions de certaines normes du code de l'urbanisme liées au littoral. Il faut souligner qu'elles sont essentielles à l'égard des spécificités de la localisation de Calais. Pour clore mon propos, je souhaite évoquer à mon tour les indemnités des marins. Vous acceptez de transposer une disposition dans la volonté d'atténuer les conséquences de la crise sanitaire due au covid-19 pour les marins. En ces termes, elle prévoit que les périodes d'activité partielle seront soumises au versement de cotisations vieillesse à compter du 1 mai 2021. Le groupe socialiste approuve bien évidemment cette mesure. Néanmoins, comme l'a souligné le rapporteur, je tiens à alerter sur un point, et non des moindres l'application de cette disposition au 1 mai 2021 va créer une discrimination par rapport aux salariés ayant débuté le chômage partiel dès le début de la pandémie, en 2020. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste réclame que la prise en compte des indemnités d'activité partielle dans le salaire de référence retenu pour le calcul de la pension des marins puisse s'appliquer dès le 1mars 2020,

ces éléments et des apports résultant de nos travaux en commission et en amont de la séance, le groupe socialiste se prononcera pour l'adoption de ce texte.

l'application du principe de subsidiarité. Ce contrôle intervient préalablement à l'incorporation de ce droit dans notre droit interne, ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Comme l'ont soulevé beaucoup de nos collègues en commission, le texte qui nous est proposé est particulièrement technique. Ce projet de loi recouvre énormément de sujets, par ailleurs très hétéroclites. Je ne pourrai évidemment pas tous les traiter dans le temps qui m'est imparti ; je me limiterai donc à évoquer seulement quelques points. Premièrement, tout comme le précédent projet de loi consacré à l'adaptation de notre droit interne au droit européen examiné l'an dernier, le Gouvernement sera habilité à légiférer par ordonnance sur plusieurs sujets. Si nous comprenons l'utilité d'avoir recours aux ordonnances dans certains cas, notamment concernant les transpositions ou les mises en conformité au droit européen, nous n'en restons pas moins vigilants. À ce titre, je salue le travail qui a été effectué concernant l'article 41 du texte. La demande d'habilitation du Gouvernement allant au-delà de ce que le droit européen propose, la restriction du champ de cette habilitation était essentielle. En tant que législateurs, il est important, surtout lorsque nous habilitons le Gouvernement, d'être clairs sur notre rôle. Deuxièmement, la question de la transposition des directives européennes en droit français est un long débat qui cristallise les passions depuis des années. Ce texte comprend douze transpositions de directives. Loin du sujet habituel de surtransposition, qui ne se justifie que lorsque notre droit est plus contraignant que celui de l'Union européenne, ce projet de loi révèle un autre problème : celui des erreurs de transposition. Nous retrouvons cet écueil dans plusieurs articles de ce texte sur les sujets environnementaux et relatifs à la biodiversité. Cela mène la France vers des mises en demeure et des procédures d'infraction que nous pourrions et devrions éviter. Il en va de même pour les retards de transposition, aussi soulevés dans ce texte. Là encore, je prône la vigilance de chacun et me réjouis des modifications apportées pour une meilleure application du droit européen, européen, dans le contexte de préparation de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne que la France assumera dans quelques mois. Le troisième point qui me paraît important concerne les mises à jour découlant du Brexit et de ses premières conséquences. Nous en vivons les effets depuis la sortie du Royaume-Uni, notamment pour ce qui concerne les transports. Je ne serais pas étonné que, dans un futur plus ou moins proche, nous devions encore adapter notre droit. Nous ne connaissons pas encore toute l'étendue des changements que la sortie d'un État membre implique pour l'Union européenne et les autres États membres. La France est en première ligne des relations post-Brexit. En tant que voisine directe de la Grande-Bretagne, elle partage beaucoup de ses valeurs. Les dernières évolutions dans nos relations ne montrent malheureusement pas une application totalement apaisée de l'accord commercial qui nous unit. De plus- et je m'exprime ici en tant que président du groupe d'amitié France-Irlande -, les événements du week-end dernier nous appellent à être attentifs au respect de l'accord, par et pour toutes les parties. De manière plus générale, ce projet de loi fixe un objectif clair : mettre à jour notre droit national en prévision de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne que la France prendra durant la première moitié de l'année 2022. C'est l'avenir de l'Europe qui sera en question. Les priorités doivent être claires. La puissance de l'Europe passe par son autonomie et sa souveraineté. Je souhaite ici dégager quelques axes qui me paraissent prioritaires à cet égard. Notre agriculture et notre alimentation doivent être placées au centre de notre souveraineté. Nous devons assumer une véritable diplomatie. Le monde pâtit beaucoup trop de l'absence d'une voix européenne unifiée et puissante. Notre politique commerciale doit évidemment évoluer et notre nouvelle stratégie doit se concrétiser afin de défendre nos valeurs et nos intérêts. Enfin, faisons de l'Europe l'un des plus grands espaces de protection de notre biodiversité. Les articles de ce texte concernant la question environnementale montrent l'importance du dossier. Le groupe Les Indépendants, très attaché aux questions européennes et à une bonne incorporation des avancées du droit européen dans notre droit interne, votera en faveur de ce projet de loi. La parole est à M. Jacques Fernique. Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues,

Sur la procédure, l'étude d'impact n'ayant été finalisée que tardivement, dans des délais restreints, il a été difficile pour le Conseil d'État d'émettre en temps utile une appréciation des mesures envisagées. Il en va de même- notre collègue Gérard Lahellec l'a déjà relevé -de certaines consultations, qui ont été effectuées dans la précipitation. Sur le fond, si l'harmonisation des régimes de responsabilité des transporteurs aériens, éventuelle d'alcool et d'autres psychotropes par les équipages ou, entre autres, l'extension de l'application des règles sur le transport aérien de matières dangereuses sont positives, le renforcement particulièrement démesuré de la répression des intrusions sur les pistes nous paraît excessif. vise des manifestations qui ne sont vraiment pas fréquentes et nous paraît relever d'un signal politique outrancier plutôt que du seul souci de sécurité.

aborder les transports terrestres et le domaine maritime. L'article 21 est évidemment positif, puisqu'il permettra d'intégrer les périodes d'activité partielle pour les droits à pension des marins.

contrairement aux mesures sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers et sur la lutte contre les pratiques abusives de cabotage, qui constituent des avancées positives. Nous sommes d'ailleurs en attente forte de la prochaine fournée du paquet mobilité.

Ces dispositions sont, on le sait, le résultat d'un travail long et très compliqué pour enfin parvenir à réprimer des pratiques qui jettent de l'huile sur ces zones de feu en contribuant

La Commission européenne a d'ailleurs mis en demeure la France pour défaut de transposition. Il était donc temps que cette mesure s'applique. Enfin, sur l'initiative de mon collègue Ronan Dantec, notre groupe a saisi l'occasion pour proposer un amendement sur un enjeu d'importance.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi que nous nous apprêtons à examiner s'inscrit dans le cadre des obligations que notre pays se doit de respecter en tant en tant qu'État membre de l'Union européenne. Il s'agit en effet d'adapter notre droit aux évolutions plus ou moins récentes de la législation européenne. Ce texte assure ainsi la transposition de pas moins de douze directives et la mise en conformité de notre droit avec quinze règlements européens, dans des domaines aussi variés que les transports, la prévention des risques, l'environnement, ou encore l'économie et les finances. Son adoption par notre Haute Assemblée est appelée à revêtir un caractère hautement symbolique alors que la France s'apprête à exercer la présidence du Conseil de l'Union européenne. En veillant à la conformité de notre droit national avec le droit européen, notre travail législatif contribuera à assurer à la France une certaine exemplarité et à lui permettre de porter plus efficacement la voix du Conseil auprès des autres organes de l'Union et de ses États membres. Dans un espace sans frontières intérieures, où les échanges sont marqués par la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, il est impératif de procéder à l'harmonisation de certaines règles, afin de garantir la sécurité des personnes, de veiller à éviter toutes formes de dumping social ou encore d'assurer la protection de l'environnement. Comme le faisait remarquer le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi, il s'agit d'un texte contenant de nombreuses mesures, complexes et spécifiques. Aussi mon intervention n'a-t-elle pas vocation à être exhaustive. Je relèverai simplement que, tout en répondant à l'impérative mise en conformité de notre droit, le texte s'ancre pleinement dans l'actualité. Certains de ses articles tirent ainsi les conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire, tandis que d'autres invitent à procéder aux ajustements rendus nécessaires par la sortie du Royaume-Uni

Germanwings en 2015, il prévoit et encadre la soumission du personnel navigant à des tests de dépistage d'alcoolémie et de substances psychoactives. Il comble également un vide en matière de transport de marchandises dangereuses par voie aérienne ; jusqu'ici, le code des transports ne prévoyait aucune disposition particulière. Le texte renforce également la sécurité des aéroports, en aggravant les sanctions encourues en cas d'intrusion illégale en zone sensible. Aujourd'hui, notre droit semble en effet beaucoup moins dissuasif que celui de la plupart des États membres. En matière de transport routier, le texte procède à la transposition de dispositions du paquet mobilité européen. Il s'agit d'une avancée considérable, puisqu'il est question de garantir aux conducteurs de véhicules lourds un socle de droits sociaux. En procédant à l'encadrement des conditions de travail des conducteurs routiers, de leur détachement, et en réglementant la pratique du cabotage, ce texte lutte en effet efficacement contre le dumping social et tend vers des conditions de concurrence plus loyale entre les opérateurs Le texte revêt également une dimension éthique en imposant aux importateurs d'étain, de tantale, de tungstène et d'or un devoir de « diligence Ces entreprises devront s'assurer par un mécanisme de conformité de la traçabilité des matières importées, tandis que les autorités compétentes devront veiller, par le biais d'un contrôle, au respect de ces obligations. qu'aucun opérateur ne cautionne par ses importations des atteintes aux droits humains ou ne finance des groupes armés non étatiques, l'Union européenne et les États qui en sont membres font bien plus que promouvoir un cadre libéral d'échanges commerciaux. Tout en assurant la promotion de leurs propres valeurs et principes, ils développent un cadre éthique pour les échanges extraeuropéens. Enfin, en abordant des sujets tels que les émissions de soufre des navires, la limitation de l'impact environnemental des activités liées au mercure, l'usage des polluants organiques persistants ou encore la pollution de l'eau, ce texte est pleinement en phase avec les préoccupations environnementales actuelles. Au moment où notre Haute Assemblée s'apprête à entamer l'étude du projet de loi Climat et résilience, il est bon de vérifier, une fois de plus, que celles-ci dépassent largement le cadre national. Elles témoignent d'une prise de conscience de dimension internationale à laquelle l'Union européenne fait écho par sa législation.

de ses politiques, plus solidaire et plus soucieuse de l'environnement. Durant sa présidence du Conseil de l'Union, la France sera en mesure de défendre cette exigence. En soutenant ce projet de loi, le groupe RDPI

C'est très éloigné des 80 % que martèlent nombre d'eurosceptiques, mais cela n'en reste pas moins substantiel ! Certains secteurs de notre législation conservent une maîtrise essentiellement, voire exclusivement nationale ; je pense à l'éducation, au logement, à l'organisation du territoire, à la justice, à la police- c'est d'actualité ! -ou encore à la défense. Mais il en est d'autres où l'Europe régule davantage, à l'image de ceux dont nous avons à discuter aujourd'hui, c'est-à-dire les transports, l'environnement ou l'économie. La discussion n'a pas toujours été de tout J'ai encore en tête les débats soutenus qui ont émaillé nos échanges autour de l'ouverture à la concurrence de notre secteur ferroviaire. On pourrait y ajouter l'agriculture, qui n'est, certes, pas notre sujet cet après-midi, mais qui est néanmoins d'actualité avec les débats en cours au sein du Conseil de l'Union européenne sur la nouvelle politique agricole commune.

-, afin de ne pas apparaître comme un mauvais élève dans la perspective de la future présidence française, qui débutera en janvier 2022. Ce sera un moment historique, puisque nous exercerons la présidence pour la première fois depuis 2009 et le traité de Lisbonne. d'une responsabilité importante, qui astreint à l'exemplarité, et d'une occasion unique, qui nous ouvrira des perspectives, pour inscrire à l'agenda européen des sujets chers à nos yeux. La préservation de notre environnement et la lutte contre le changement climatique en font indéniablement partie et ne sont- fort heureusement ! -pas absents du présent projet de loi.

parle pas du retard important qui a été pris pour la mise en conformité de notre droit. C'est en particulier le cas en matière de protection de l'environnement, avec les réglementations sur le mercure et les fluides frigorigènes, ou sur la préservation des espèces animales protégées : la France a reçu une mise en demeure pour non-respect de cette directive adoptée voilà près de trente en 1992 ! Cette mise en conformité tardive fait malheureusement écho aux propos que je tenais ici même la semaine dernière, lors du débat sur le projet de loi constitutionnelle. Gageons que ce projet de loi de transposition sera l'une des nombreuses pierres qu'il nous faudra assembler dans les prochaines années si nous souhaitons être dignes des engagements pris ici ou dans le cadre de l'accord de Paris. Notre groupe défendra d'ailleurs un amendement visant à renforcer notre droit en matière d'évaluation des conséquences sur l'environnement de certains projets publics ou privés, dans la droite ligne de l'esprit de la directive de 2011 ou de la décision rendue le mois dernier par le Conseil d'État. Au-delà de l'environnement, le texte contient des dispositions sensibles et décline des aménagements rendus impératifs par le Brexit, afin notamment de préserver les intérêts de nos entreprises, qu'il s'agisse de l'accompagnement des pêcheurs, durement touchés par la crise du coronavirus, ou de la préservation des intérêts de nos compagnies de transport maritime. enfin le travail fourni par notre commission, saisie au fond sur trente et un des quarante-deux articles que comporte le texte. Plusieurs modifications ont été apportées, avec l'objectif de renforcer encore les garanties de conformité de notre droit aux prescriptions de l'Union européenne, comme en matière de teneur en soufre des combustibles marins ou de droit de pause des travailleurs mineurs effectuant un stage à bord de navires, une disposition supprimée de notre droit par erreur en 2010.

Enfin, je me réjouis de l'ouverture aux collectivités territoriales de la possibilité d'obtenir une délégation de l'État pour l'organisation des lignes d'aménagement du territoire en direction d'autres pays membres de l'Union européenne. Cette préconisation est issue de la mission d'information du Sénat sur les transports aériens, dont notre ancienne collègue Josiane Costes était rapporteure. La mise en conformité de notre droit avec les réglementations européennes est une obligation. Faisons en sorte qu'elle soit aussi une occasion d'aller plus loin et d'être plus efficace. Notre groupe se prononcera en faveur de ce texte. La parole

Le champ du présent texte est si large- il va de l'usage des drones à la lutte contre la pollution au mercure, en passant par le télépéage ou les minerais de conflits -qu'il me serait impossible de l'appréhender dans son entièreté, surtout dans le temps limité qui m'est imparti. Ce serait d'ailleurs inutile, puisque nos rapporteurs l'ont très bien fait. J'en profite pour les féliciter de la qualité de leur travail, surtout face à un texte aussi touffu et technique. Et je ne résiste pas au plaisir de constater qu'avec deux rapporteurs sur trois, mon groupe, l'Union Centriste, est particulièrement bien représenté.

accompagner la transition environnementale mise en oeuvre dans notre pays à l'échelle de l'Union européenne. C'est sur ce dernier point que je vais maintenant me concentrer. Le transport est, avec la production d'énergie, la question centrale de la transition environnementale. ce secteur représente, hors émissions importées, environ 40 % des émissions françaises et européennes de gaz à effet de serre. Dans ces conditions, nul ne saurait plus douter de la nécessité de verdir nos déplacements. Pour ce faire, la relance du fret ferroviaire est une clé incontournable. Ce dernier a été littéralement abandonné depuis quarante ans. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le réseau autoroutier a plus que doublé depuis 1980, passant de 4 900 kilomètres à 11 000 que, dans le même temps, le réseau ferré national a régressé, passant de 34 000 kilomètres à 29 000 kilomètres. La part modale du fret ferroviaire a été divisée par trois depuis 1985, époque à laquelle celui-ci représentait 30 % du transport de marchandises

Mais, à la seule échelle nationale, de telles mesures seront impuissantes à faire bouger les lignes en faveur du fret ferroviaire, car elles ne feront que contribuer à pénaliser les opérateurs nationaux, au bénéfice des transporteurs étrangers, c'est-à-dire de ceux qui achètent leur carburant hors de nos frontières et gonflent leurs réservoirs pour ne pas avoir à se ravitailler en France. La solution ne peut être qu'européenne. C'est d'ailleurs la même problématique que l'on retrouve dans le domaine du transport aérien. aérien. Interdire les vols intérieurs courts va inévitablement conduire à un report modal vers les aéroports d'autres villes européennes pour les vols de correspondances, avec un bilan carbone plus lourd. Là encore, c'est à l'échelle de l'Union européenne que les choses se jouent. Par-delà les aménagements nécessaires de notre droit que le présent texte opère, le verdissement de notre pays passera donc par celui des transports européens. Or ce dernier n'est pas assuré. Par exemple, la directive Eurovignette est en panne.

Mon propos s'inscrira dans le prolongement de celui de notre rapporteur, Cyril Pellevat, dont je salue le travail. Avant de passer en revue les dispositions qui doivent attirer notre attention, je vais dévoiler notre position : mon groupe politique votera pour l'adoption de ce projet de loi.

même pour l'article 10 sur les sanctions applicables dans le droit français pour punir l'intrusion en zone « côté piste » d'un aéroport. La position de fermeté de notre rapporteur sur ce point est, je le crois, le meilleur choix. autre disposition dont on peut saluer l'élaboration. Il transpose la directive du 19 mars 2020 sur les systèmes de télépéage routier. Mais deux axes doivent également retenir l'attention du législateur. Il y a d'abord les dispositions afférentes « travail à la pêche ». La première, l'article 20, porte sur le travail de nuit des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à bord des navires. Par cohérence, lisibilité et volonté de respecter l'article 12 de la directive 94/33/CE, la commission a souhaité réintroduire dans le droit national des dispositions garantissant un temps de pause aux jeunes aux jeunes travailleurs à bord des navires de pêche. La modification était bienvenue. La deuxième, l'article 21, porte sur la prise en compte des périodes d'activité partielle pour la validation des droits à pension des marins. À l'instar de notre collègue Cyril Pellevat dans son rapport, je regrette que le Gouvernement que le Gouvernement ne soit pas allé plus loin dans sa volonté de sécuriser les droits sociaux des marins. M. le rapporteur souligne : « [ ...] soumettre rétroactivement à cotisation les périodes d'activité partielle sur une période plus longue aurait pour conséquence de permettre des surclassements supplémentaires, ce qui induirait indirectement des droits à pension plus élevés dans le futur. » D'où une irrecevabilité au titre de l'article 40 de la Constitution. En d'autres termes, si le Sénat n'ignore pas la nécessité de sécuriser les droits sociaux des marins, il ne lui revient pas de légiférer en ce sens. Chacun comprendra à qui cette responsabilité incombe incombe ... Je souhaite également évoquer la transposition du paquet mobilité I aux articles 22 et 23. Ces dispositions sont sans doute les plus « politiques » du texte. La réforme du paquet mobilité est ambitieuse. Elle s'attaque à plusieurs défis : le détachement des chauffeurs routiers, le temps de repos ou encore la limitation du cabotage. C'est une parfaite illustration des difficultés que pose la construction européenne, mais aussi des moyens pour les surmonter. Après trois ans de négociations, négociations qui n'étaient pas seulement déterminées par une opposition entre l'Est et l'Ouest, nous avons pu obtenir un accord, certes imparfait, mais qui sera un nouvel outil pour lutter contre la concurrence déloyale et le dumping social, sur lequel certains de nos partenaires européens prospèrent. Le projet de loi va ainsi permettre de lutter contre le cabotage systématique en introduisant une période de carence de quatre jours avant que d'autres opérations puissent être effectuées dans le même pays avec le même véhicule. Une autre mesure, moins concrète, mais sans doute plus décisive à long terme est la transposition de l'article 1

en établissant qu'il s'applique aux opérations de cabotage, mais pas aux parcours de transit. Je voudrais m'arrêter sur un dernier point. L'article 32 vise à mettre en conformité le droit national avec le droit européen concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, à la suite de la procédure d'infraction pour non-conformité lancée par la Commission européenne. Aujourd'hui, en droit français, une information doit, pour être qualifiée d'environnementale, avoir « pour objet » les éléments mentionnés à l'article L. 124-2 du code de l'environnement, alors que la directive définit l'information environnementale comme toute information disponible « concernant » ces éléments. L'article vise donc à consacrer une définition de l'information environnementale identique à celle de la directive. Mesure-t-on les conséquences d'une telle modification ? L'étude d'impact nous précise qu'il s'agit de « lever toute ambiguïté sur ces points ». Espérons en effet qu'il ne s'agisse que de clarification rédactionnelle ! Pour conclure, malgré quelques interrogations, fondées je le crois, il n'y a rien dans ce projet de loi qui puisse compromettre son adoption. La parole

Mon intervention porte donc sur un point très précis du présent projet de loi, mais ô combien important. Comme tous les textes d'adaptation au droit de l'Union européenne, celui qui nous est soumis aujourd'hui embrasse un large champ. Et au milieu de tout cela, on trouve l'article 24, un OLNI : objet législatif non identifié ! Cet article est aussi lapidaire qu'insatisfaisant. Sa clarté est inversement proportionnelle à l'importance de son enjeu. Cet enjeu, quel est-il ? Au mois de juin dernier, dans le cadre du Brexit, le Gouvernement a demandé à Eurotunnel, comme aux ports maritimes, de construire des infrastructures destinées à accueillir les services assurant les contrôles douaniers et sanitaires aux frontières. En effet, le Royaume-Uni devenant un pays tiers par rapport à l'Union européenne, il fallait rétablir ces contrôles, qui se traduisaient par la réalisation de bâtiments et la mise en oeuvre des moyens matériels correspondants. Eurotunnel s'est immédiatement exécuté. Compte tenu de l'urgence, ces travaux ne pouvaient pas satisfaire aux autorisations d'urbanisme. C'est pourquoi, par son ordonnance du 24 janvier 2019, le Gouvernement a dispensé Eurotunnel de ces formalités pour procéder aux aménagements demandés. L'autorisation était temporaire et la situation devait encore être régularisée, cette fois non pas par ordonnance, mais par une disposition législative destinée à assurer la pérennité des infrastructures. Cette disposition législative, c'est l'article 24 du présent projet de loi, qui est triplement insatisfaisant. Premièrement, d'un point de vue formel, sa rédaction était clairement obscure, puisque le nom du code de référence, à savoir le code de l'urbanisme, n'y figurait pas. Je remercie notre rapporteur, Cyril Pellevat, d'avoir corrigé ce regrettable oubli. Deuxièmement, sur le fond, on ne comprend pas si cet article valide seulement les infrastructures déjà réalisées par Eurotunnel ou s'il conforte les aménagements qui devront encore être réalisés. Si tel n'est pas le cas, faudra-t-il obtenir à chaque fois une autorisation législative spécifique ? Ce serait tout de même kafkaïen ! L'article fait de plus peser sur Eurotunnel une vraie insécurité. Les aménagements liés à la sécurité, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires à son fonctionnement ne sont pas possibles. Croyez-vous sincèrement que le tunnel ne soit pas concerné ? Il l'est au premier rang. Troisièmement, et de manière bien plus fondamentale, le problème ponctuel du Brexit et des aménagements douaniers soulève la question du statut juridique du tunnel sous la Manche. Le tunnel n'est à l'évidence pas une simple ligne ferroviaire. Cette infrastructure est exceptionnelle ; il serait temps de la considérer comme telle. Des navettes transportent des camions, des voitures particulières, des bus sur une ligne prédéfinie.

Aujourd'hui assimilé à une infrastructure ferroviaire simple, ses marges de manoeuvre sont d'autant plus restreintes que l'ouvrage ne figure pas aux exceptions de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, contrairement aux ports et aux aéroports. C'est cela qu'il faut changer. La question est : quelle est notre ambition pour cet ouvrage unique au monde, clé pour le développement national et vital à l'échelle locale ?

provoqué par le suicide d'un pilote, l'Union européenne a décidé d'imposer des tests de dépistage d'alcool et de substances psychoactives au personnel du transport

a néanmoins souligné que la mise en oeuvre du dispositif de contrôle devait s'effectuer dans le respect du secret médical, notamment afin de préserver la vie privée des

En pratique, les tests d'alcoolémie sont fiables, et le doute concerne essentiellement le cas de substances psychoactives prescrites par un médecin. C'est surtout dans cette hypothèse que les personnels redoutent les « faux positifs ». L'article 1 prévoyant une habilitation à légiférer par ordonnance, nos interrogations sur les modalités

fixer un cadre plus clair avant de confier de nouvelles compétences de régulation à une autorité indépendante. Nous pourrions courir un risque à changer ainsi les règles, alors que l'État lui-même a confié

mois. Conformément au principe d'indépendance régissant l'exercice par l'ART de ses missions, l'ordonnance n° 2019-761 du 24 juillet 2019 avait pris soin d'ériger au rang législatif les missions de l'Autorité en matière de régulation aéroportuaire. Il nous semble important de permettre à l'ART de notifier les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et de les rendre publics, pour une question de transparence. Il apparaît

n° 7 rectifié a pour objet de lever toute ambiguïté sur le champ du pouvoir réglementaire reconnu à l'ART concernant les principes d'allocation des actifs, produits et charges.

l'avis de la commission ? Avec huit amendements déposés sur l'article 6, le thème de la régulation aéroportuaire par l'Autorité de régulation des transports est un sujet important de notre débat en séance publique.

Faut-il pour autant modifier cet équilibre ? La régulation repose sur un socle de transparence et de concertation préalable entre tous les acteurs. Or, dans le temps qui nous a été imparti pour examiner ce texte, nous avons vu apparaître des divergences entre le régulateur, l'État et les opérateurs.

en particulier sur sa différence de point de vue avec le régulateur, sur l'équilibre des relations entre les aéroports et les compagnies aériennes et sur l'intérêt des usagers. Le présent amendement prévoit de donner à l'ART la possibilité de fixer les modalités d'application du principe de répartition entre le secteur régulé et le secteur non régulé.

Cet amendement vise à préciser le périmètre de la collecte d'informations prévue par le texte de la commission pour permettre au régulateur d'accomplir sa mission dans le domaine aéroportuaire. Quel est l'avis

à l'Autorité de régulation des transports une mission de suivi économique et financier des aérodromes entrant dans son champ de compétence, ainsi qu'une mission d'information de l'ensemble des acteurs du secteur. L'efficacité de la régulation implique que tous les acteurs, notamment les compagnies aériennes et leurs représentants, disposent d'informations objectives et agrégées sur la situation économique et financière des aéroports. Il nous semble donc indispensable de compléter cet article 6 pour confier à l'ART,

de la commission ? Ces amendements visent à renforcer le suivi économique et financier des aéroports par l'Autorité de régulation des transports. Il s'agit d'une extension des pouvoirs de l'ART qui dispose, ponctuellement, pour réaliser ses missions, de pouvoirs d'investigation. D'un point de vue rédactionnel, l'amendement renvoie à l'article L. 1264-2 du code des transports, qui donne des pouvoirs d'information étendus au régulateur dans le domaine ferroviaire. Cet article assez volumineux se compose de de douze alinéas et prévoit un droit d'accès à la comptabilité des opérateurs, un large droit à l'information auprès des entreprises intervenant dans le secteur ferroviaire, des pouvoirs d'enquête, le recours à des audits, etc. On peut donc s'interroger sur la rédaction retenue, car la base législative prise comme référence porte assez spécifiquement sur le secteur ferroviaire. C'est pourquoi je propose de recueillir la position du Gouvernement pour aboutir à une solution consensuelle. La commission s'en remet à la sagesse

de la commission ? Cet amendement vise à supprimer l'article 9, au motif que ce texte n'est pas le bon vecteur législatif pour en discuter. Il est vrai que, en matière de sécurité des transports, le ferroviaire et la RATP ont été traités dans la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, un texte définitivement adopté et en cours d'examen par le Conseil constitutionnel. Cependant, à la différence de ces deux modes de transports, le transport aérien a une dimension beaucoup plus internationale. C'est pourquoi il est très largement régi par le droit européen. En l'occurrence, deux règlements européens récents- (UE) n° 2019/103 et (UE) n° 2019/1583 -étendent à de nouvelles catégories de personnels intervenant dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile les obligations d'effectuer une vérification de leurs antécédents. L'article 9 n'est ici que le prolongement des engagements de la France visant à renforcer la sécurité aérienne.

est pas moins nécessaire de mettre en conformité le droit national avec le droit de l'Union européenne dans le domaine de la sûreté aéroportuaire. Cet ensemble de mesures vise à prévenir les actes malveillants contre l'aviation civile.

et attentatoires aux initiatives citoyennes : point n'est besoin d'être si liberticide ! Nos plateformes et nos avions ne sont pas si menacés que cela.

Or les zones à protéger sont vastes. Il faudrait déployer des bataillons de forces de sécurité en dégarnissant d'autres zones sensibles de notre territoire ; ce n'est pas ce que je préconise. Troisièmement, on constate que les sanctions envisagées à cet article pour l'aéroportuaire correspondent à celles qui sont prévues pour les intrusions sans autorisation dans une zone d'accès restreint d'un port. On peut également signaler que les sanctions proposées- six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende -pour protéger les zones sensibles portuaires et aéroportuaires représentent la moitié des sanctions prévues en cas d'intrusion non autorisée dans l'emprise d'installations nucléaires.

12, 13 et 14 de l'article 13 confient à l'ART une mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage. Il nous paraît plus pertinent de limiter le périmètre de la mission de conciliation qui serait confiée à l'ART à la vérification, d'une part, que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage

l'avis de la commission ? Il nous semble que la directive est imprécise quant au champ exact des compétences de l'organe de conciliation. L'adoption de ces amendements permettrait d'éviter toute ambiguïté. En outre, leurs dispositions me semblent conformes à la directive européenne, qui mentionne, dans son considérant 30, que l'organe de conciliation est compétent pour s'assurer du « caractère non discriminatoire

que les conditions contractuelles appliquées aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et que ses prestataires sont rémunérés sur des bases équitables. Toutefois, l'usage même des mots « en particulier » implique que la mission de conciliation entre percepteurs de péage et prestataires du service européen de télépéage ne se limite pas à ces deux sujets on pense notamment à la non-discrimination et aux conditions de rémunération. Pour rappel, l'article 10 de la décision 2009/750/CE prise par la Commission pour les besoins de l'application de la précédente directive Télépéage prévoyait déjà qu'un organe soit chargé d'une mission de conciliation entre percepteurs de péage et prestataires du service. Il le faisait en des termes quasi identiques à ceux de l'article 11 de la nouvelle directive. Or le décret n° 2012-645 du 3 mai 2012 organisant une commission de conciliation du télépéage, abrogé en 2020 à des fins de simplification administrative, avait transposé cet article 10 de manière similaire. La rédaction proposée à l'article 13 du présent texte permet La rédaction proposée à l'article 13 du présent texte permet donc de conserver une cohérence dans la transposition des textes communautaires relatifs au télépéage tout en évitant cette sous-transposition, qui ne semble pas souhaitable. J'émets donc un avis défavorable.

Il nous paraît plus pertinent que cette mission d'enregistrement reste exercée par ce ministre ou, à défaut, qu'elle le soit par une autre entité administrative compétente en la matière.

La mission consistant à vérifier que ces prestataires remplissent les conditions requises par la réglementation, notamment qu'ils disposent des capacités techniques, financières et

afin de limiter les effets nocifs des oxydes de soufre sur l'environnement et sur la santé humaine. Depuis le 1 janvier 2020, la teneur en soufre des combustibles utilisés par les navires en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre est fixée à 0,50 Un amendement à la convention Marpol est entré en vigueur le 1 mars 2020. Il complète ce dispositif en interdisant également le transport, aux fins de combustion, de combustibles dont la teneur en soufre est supérieure à 0,50 %, à moins que le navire ne soit équipé d'un dispositif d'épuration des gaz d'échappement approuvé par les autorités. Il s'agit d'une mesure additionnelle visant à renforcer l'effectivité et l'application uniforme des plafonds de teneur en soufre. Ces dispositions n'ayant pas encore été transposées dans le droit national, j'émets un avis très favorable sur cet amendement. Quel est l'avis du Gouvernement ? Dès lors Gouvernement ? Dès lors que ces navires ne sont pas équipés d'un dispositif permettant de réduire les émissions, le seuil est effectivement fixé à 0,5 % de la masse par la convention Marpol. La limitation de la teneur en soufre est reprise par la directive européenne 2016/802, dont l'article 16 du présent texte parachève la transposition. La règle du, adoptée par l'Organisation maritime internationale, est entrée en vigueur le 1 mars 2020.

nous abordons le cas des jeunes marins, que j'ai évoqué dans mon intervention liminaire.

est l'avis de la commission ? La rédaction du projet de loi initial vise à prendre en compte la réalité du travail dans le secteur maritime. En son état actuel, le droit ne permet pas toujours aux jeunes qui effectuent des stages à bord de navires d'embarquer, l'embarquement ayant généralement lieu avant cinq heures du matin. Il apparaît nécessaire de remédier à cette situation pour favoriser l'employabilité des jeunes et leur permettre de découvrir les métiers maritimes. La commission a donc émis un avis défavorable. Par ailleurs, je tiens à rappeler que la mesure ne concerne que les jeunes âgés d'au moins 16 ans et qu'elle est strictement conforme à la directive 94/33/CE, laquelle n'impose un repos obligatoire qu'entre minuit et quatre heures du matin. Au cours des auditions en Au cours des auditions en commission, j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs organisations professionnelles de gens de mer. Elles n'ont pas fait état d'inquiétudes sur ce point. Au contraire, elles ont mentionné l'utilité de cette mesure pour tenir compte des horaires et contraintes des métiers maritimes et permettre aux jeunes de découvrir la vie d'un navire lors de leurs stages.

nous transposerions une forme de droit opposable à une revendication considérée comme légitime, ce qui poserait quand même un petit problème de fond.

et le trafic transmanche va subir des turbulences supplémentaires en raison du Brexit. La France est un grand pays maritime, à la façade développée. Il importe que les compagnies puissent continuer leur activité en employant le plus de marins français afin de maintenir l'emploi et le savoir-faire marin sur notre territoire c'est un impératif de souveraineté. Or la compétitivité de ces entreprises est menacée. Avec cet amendement, nous proposons des exonérations de cotisations afin de soutenir ce secteur vital face aux crises qui le frappent et d'en améliorer la compétitivité.

Lors de mes travaux, des représentants du secteur maritime m'ont fait part de leurs inquiétudes à ce sujet. Toutefois, l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit déjà une exonération de cotisations et de contributions sociales pour le transport maritime de passagers jusqu'au 31 décembre 2021. De plus, le PLFR 4 a prévu pour les entreprises de transport de passagers soumises à la concurrence internationale une aide à hauteur de 30 millions d'euros à travers le remboursement de la part salariale des cotisations sociales en 2021. Enfin, le décret mettant en place un dans le secteur maritime vient d'être publié. Il prévoit des exonérations de cotisations personnelles et de contributions sociales pour les compagnies maritimes effectuant des trajets internationaux.

Madame la secrétaire d'État, prévoyez-vous d'autres mesures pour venir en aide aux compagnies de ferries, notamment à Brittany Ferries, qui est, je le rappelle, le premier employeur de marins en France et qui connaît des difficultés dramatiques ? Il sera également nécessaire de débattre de la pérennisation de ces dispositifs dans le cadre des négociations du Fontenoy du maritime. Quel est l'avis du Gouvernement

Je tiens à intervenir sur la question extrêmement sensible du travail détaché dans le domaine du transport de marchandises. Ce matin, en commission,

Comment, au nom de la liberté de circulation, notre Europe a-t-elle pu permettre une telle déstructuration du secteur du transport de marchandises ?

s'était engagé en 2017 à régler vite la question du travail détaché. Lors de l'une de ses premières sorties à Bruxelles, il avait obtenu des progrès pour bien des secteurs- je tiens à le signaler -, mais pas pour le transport de marchandises. Il a fallu attendre le paquet mobilité et l'action résolue du Parlement européen européen pour obtenir ces décisions, que nous allons voter, car elles constituent un progrès significatif. Je tiens à signaler le rôle de la présidente de la commission des transports et du tourisme

Il était prévu que les dispositions puissent être communiquées aux partenaires sociaux ; nous proposons qu'elles soient communiquées aux organisations syndicales et patronales afin que celles-ci aient accès à toute l'information. Quel est l'avis de la commission ? L'alinéa 32 de l'article 23, dans sa rédaction actuelle, prévoit la possibilité de communiquer aux partenaires sociaux certaines informations disponibles dans le système d'information du marché intérieur permettant de vérifier le respect des règles en matière de détachement qui seront fixées par voie réglementaire. Cela me semble conforme à la directive, laquelle prévoit bien une faculté et non une obligation. L'adoption de cet amendement permettrait de clarifier la rédaction actuelle et pourrait garantir une application plus rigoureuse et transparente des règles du détachement.

soient communiquées aux organisations syndicales et patronales représentatives dans les branches professionnelles concernées. Cette précision me semble tout à fait cohérente avec les objectifs de la disposition, même si l'on pourrait considérer qu'elle relève du niveau réglementaire. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.

Ainsi que je l'ai évoqué dans la discussion générale, cet amendement vise à réécrire l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme afin de rétablir une égalité de droits entre les ports, les aérodromes et la liaison fixe transmanche. La rédaction en vigueur dudit article ne mentionne pas la liaison fixe, qui se trouve dès lors exclue du régime dérogatoire octroyé aux ports et aux aérodromes. L'article 24 du projet de loi limite la régularisation des installations de la liaison fixe aux seules « installations, constructions et aménagements nécessaires

des camions, avec du fret, des véhicules de tourisme, des bus et elle permet, parallèlement, le passage direct de l'Eurostar. Pourquoi donc faire une différence ? Pourquoi ne pas profiter de cet événement pour lever cette incertitude et répondre à cette

du droit, il me semble que, en l'espèce, la codification n'est pas opportune, compte tenu de la nature des dispositions. En effet, l'article 24 a un objet très strict : il vise uniquement à régulariser les installations construites au niveau du lien fixe transmanche pour tenir compte du rétablissement des contrôles à la suite du Brexit. En pratique, il s'agit donc uniquement de permettre la délivrance d'un permis de construire et en aucun cas de créer des possibilités d'aménagements futurs. Deuxièmement, sur le fond, cet amendement vise à introduire une dérogation à la loi Littoral au bénéfice du site Eurotunnel. Je n'y suis pas favorable pour trois raisons.

Toutefois, il s'agissait de permettre la densification d'espaces creux situés dans des zones déjà urbanisées. L'atteinte portée à la loi Littoral et au principe d'urbanisation en continuité des constructions existantes était donc limitée. La loi Littoral repose sur la recherche d'un équilibre entre les impératifs de protection de l'environnement et d'aménagement. Il me semble que, en l'espèce, l'équilibre proposé par l'amendement n'est pas satisfaisant. Ensuite, si je comprends les enjeux économiques soulevés en matière de concurrence entre les modes de transport, il me semble difficile de mettre les ports, comme le port de Calais, et Eurotunnel sur le même plan en matière de préservation du littoral, dans la mesure où ils ne sont pas soumis au même statut juridique. Les ports relèvent du domaine public. Autrement dit, les autorités publiques disposent d'un moyen de contrôle des décisions d'aménagement qui y sont prises. Ce n'est pas le cas d'Eurotunnel, qui est une entité privée. Si nous introduisions une dérogation à la loi Littoral pour le lien transmanche, nous exposerions potentiellement une zone littorale sensible à un risque d'étalement des constructions en dehors de tout contrôle de l'État. Cela ne me semble pas souhaitable. Enfin, je tiens à souligner que le terminal d'Eurotunnel et les installations connexes sont situés à la limite des communes de Coquelles et de Fréthun,

introduire une telle dérogation dans le code de l'urbanisme porterait une atteinte à la loi Littoral qui me semble disproportionnée. La question soulevée par cet amendement est toutefois intéressante : d'après les éléments que j'ai pu rassembler, Eurotunnel risque de faire face à des besoins nouveaux en matière d'aménagement dans un futur proche, notamment en raison de l'entrée en vigueur de la réglementation européenne,

dont bénéficient déjà les installations nécessaires au fonctionnement des services publics portuaires. Nous avons dû permettre à Eurotunnel de déposer un permis de construire de régularisation des infrastructures de contrôles frontaliers existantes. Il fallait régulariser des installations déjà construites, dans le contexte que l'on connaît, mais surtout pas étendre de manière pérenne cette dérogation,

M. Jean-Pierre Corbisez. Deux lettres de mise en demeure ont été adressées à la France par la Commission européenne portant sur les lacunes de la législation française transposant la directive Projets de 2011 sur deux points l'obligation de prendre en considération l'ensemble des critères établis en annexe III de la directive pour déterminer si un projet doit être soumis à évaluation environnementale ; l'obligation de veiller à ce que les autorités compétentes accomplissent leur mission de manière objective. La nomenclature des projets soumis à évaluation a été annulée par le Conseil d'État le 15 avril dernier, au motif qu'elle se fonde essentiellement sur la dimension du projet. Quant à la prévention des conflits d'intérêts, le décret du 3 juillet 2020, qui organise un système de déport, ne semble pas non plus suffire à la Commission.

comme le proposent nos collègues du groupe écologiste par un amendement que nous avions cosigné par le passé. La seconde issue, que nous vous soumettons par cet amendement, est de supprimer les critères et les seuils définis par voie réglementaire et de laisser l'autorité environnementale indépendante décider au cas par cas de soumettre, ou non, le projet à évaluation environnementale, en se fondant sur les termes de la directive. Tant que l'autorisation du projet et l'examen au cas par cas relèveront de la même autorité, les contentieux devant les tribunaux administratifs perdureront. Le Conseil d'État a rappelé, dans un arrêt du 28 avril 2021, que l'autorité environnementale doit disposer d'une autonomie réelle et, à ce titre, être pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres. Confier à un préfet de région le soin, à la fois, de décider de l'opportunité de mener l'évaluation et d'autoriser le projet constitue une violation du principe de séparation fonctionnelle et un vice de procédure substantiel. cet amendement aurait également pour avantage de simplifier la procédure en amont de l'évaluation environnementale pour le maître d'ouvrage. Il nous semble qu'une remise à plat de la législation est indispensable et préférable aux divers raccommodages intervenus en réaction à la jurisprudence du Conseil d'État.

répondre à votre proposition de supprimer totalement l'utilisation de critères et de seuils pour déterminer quels projets sont soumis à étude d'impact environnementale, afin de généraliser la méthode du cas par cas. À cet égard, je souhaite exprimer trois réserves. Premièrement, cette proposition va au-delà, à la fois, de la mise en demeure adressée à la France et de l'injonction prononcée par le Conseil d'État. La Commission européenne n'appelle pas la France à généraliser la méthode du cas par cas. Elle se borne à l'inviter à mieux prendre en compte les critères établis à l'annexe III de la directive 2011/92/UE pour « déterminer si un projet relatif à une installation doit faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement », parmi lesquels les caractéristiques du projet et sa localisation. Or ces critères sont déjà pris en compte au niveau législatif, à l'article L. 122-1, qui prévoit que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par « leur nature, leur dimension ou leur localisation » font l'objet d'une évaluation. Le problème se situe, à mon sens, plutôt au niveau réglementaire, l'article R. 122-2 du code de l'environnement exemptant de toute évaluation environnementale certains projets sur la base de critères purement quantitatifs, sans prendre en compte leurs caractéristiques et leur localisation, comme le prévoit la partie législative du code. Le Conseil d'État ne dit d'ailleurs pas autre chose dans sa décision du 15 avril dernier : il invite le Gouvernement à se mettre en conformité avec la directive, en prenant des « mesures réglementaires » permettant la soumission à évaluation environnementale de projets pour des critères autres que quantitatifs, notamment leur localisation. Deuxièmement, il me semble que votre proposition pourrait engendrer un alourdissement de procédure significatif au niveau local, puisque tout projet pourrait être soumis à étude d'impact au cas par cas. Il me semble, mais j'aimerais entendre l'avis du Gouvernement sur ce point, que cette généralisation de la méthode du cas par cas est susceptible d'induire une charge de travail sensiblement accrue pour les préfectures de région en termes d'instruction des dossiers, puisque l'autorité compétente devra potentiellement évaluer l'opportunité d'une étude d'impact pour chaque projet. je ne suis pas certain que la généralisation de la méthode du cas par cas aille dans le sens d'un renforcement de l'évaluation environnementale, puisque vous supprimez le principe d'une soumission systématique à étude d'impact pour de nombreux projets, notamment les projets de grande taille. J'en viens au deuxième point de l'amendement, qui vise à garantir une meilleure séparation fonctionnelle entre l'autorité chargée d'autoriser le projet- le préfet de région - et l'autorité chargée d'effectuer l'évaluation environnementale, qui est incarnée par les missions régionales d'autorité environnementale au niveau local depuis la loi de 2019 relative à l'énergie et au climat. Ce point est effectivement soulevé par la mise en demeure prononcée par la Commission européenne, qui mentionne des risques de conflit d'intérêts. Je souhaite toutefois entendre l'avis du Gouvernement sur la rédaction proposée et sur la manière dont il entend donner suite à la mise en demeure adressée à la France sur ce sujet. En attendant, l'avis de la commission est défavorable.

Comme indiqué à l'instant, je souhaite entendre l'avis du Gouvernement sur la rédaction proposée et sur les conséquences qu'il prévoit de tirer de la mise en demeure prononcée à l'encontre de la France. Je me prononcerai en fonction de cet avis. Enfin, l'amendement n° 5 rectifié de M. Dantec cet avis. Enfin, l'amendement n° 5 rectifié de M. Dantec soulève un sujet intéressant, qui a d'ailleurs été évoqué à plusieurs reprises au Sénat ces dernières années. Toutefois, je me dois d'exprimer plusieurs réserves. D'une part, les conséquences juridiques à tirer de la décision du 15 avril 2021 du Conseil d'État mériteraient un examen plus approfondi. Le Conseil d'État n'appelle pas le législateur à intervenir, mais invite le Gouvernement à prendre des « mesures réglementaires » afin de se mettre en conformité avec la directive européenne 2011/92/CE. Il semble donc qu'une mesure réglementaire pourrait être suffisante. J'ai bien entendu toutefois l'appel de M. Dantec. D'autre part, le Conseil d'État n'appelle pas à l'introduction d'une clause de rattrapage, mais simplement à ne pas instaurer de seuils qui auraient pour effet d'exempter totalement d'évaluation environnementale des projets qui, du fait de leurs caractéristiques ou de leur localisation, pourraient avoir des incidences négatives sur l'environnement. Enfin, je m'inquiète des conséquences de l'introduction d'une telle clause en droit français à deux titres. Premièrement, il me semble qu'elle pourrait porter atteinte à la sécurité juridique des projets déjà autorisés, puisque tout projet pourrait faire l'objet d'une procédure de rattrapage. Deuxièmement, la mesure proposée pourrait être très lourde pour certains petits projets, notamment dans le domaine agricole.

de l'autorité environnementale a été conforté par des arrêts récents du Conseil d'État. Celui-ci a jugé que, en application du droit européen, ces fonctions d'autorité décisionnaire et d'autorité chargée de l'examen au cas par cas

en deçà des seuils ne relève pas de la compétence du législateur, mais est d'ordre réglementaire. C'est d'ailleurs à cette fin que le Conseil d'État a enjoint au pouvoir réglementaire de la mettre en place. L'avis est donc défavorable sur ces trois

soit une augmentation de 276 % par rapport à 2015, première année pleine d'application de la réglementation française sur ce mode de financement. Nous voyons bien que le financement participatif se développe de manière importante et qu'il est essentiel dans différents secteurs, comme la culture, le social, l'associatif

Dans cette optique, et afin d'enrichir le débat, la commission des finances a apporté des compléments importants dans la mise en oeuvre de cet article 41, notamment pour élargir ces financements aux projets des collectivités, quelle que soit leur nature. Un tel élargissement est particulièrement pertinent à l'heure de la mise en oeuvre de la transition écologique. Au-delà, le Gouvernement ne devrait-il pas mener une réflexion d'ensemble à ce sujet, afin d'éviter tout risque de morcellement des dispositions déjà existantes ? Le financement participatif mérite en effet une attention toute particulière.

le paragraphe introduit en commission, car il n'apporte, en l'état de la réflexion, qu'une réponse incomplète aux souhaits de modification de la réglementation. Tout d'abord, il convient de rappeler que le financement participatif sous forme de prêts et de dons est déjà ouvert aux collectivités territoriales, pour tout service public. En revanche, il est exact d'affirmer que, pour sécuriser le maniement de fonds publics induits, la règle veut que le financement participatif soit réalisé une régie de recettes. Par exception, le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 a ouvert la possibilité à un tiers, une plateforme en l'occurrence, de collecter des fonds hors régie de recettes, par la voie du financement participatif, et ce quels que soient l'objet du financement et le mode de financement utilisé, y compris la levée obligataire. constituerait une dérogation totale, qui viderait de son sens le principe selon lequel une régie de recettes doit être constituée. Or ce principe doit, selon moi, être préservé pour assurer le bon maniement des deniers publics. Le recours au financement participatif par les collectivités territoriales répond, en général, au souhait de financer des projets symboliques, à forte composante extrafinancière. Par conséquent, il est proposé de circonscrire l'ouverture du périmètre de la dérogation à la régie de recettes aux champs véritablement susceptibles de bénéficier d'un financement de projet, à savoir les services publics culturel, éducatif, social et solidaire, ainsi que la protection de l'environnement, le sport et tourisme.

ne comporte pas de garde-fous qui garantiraient le développement du financement participatif de manière sécurisée. En effet, l'élargissement du recours au financement participatif se double de risques possiblement accrus de collusion de faits susceptibles d'entraîner une qualification pénale. Aussi, le Gouvernement propose de renforcer les sauvegardes et de préciser les obligations des plateformes, appliquées au financement des projets des collectivités territoriales. Tel est, l'objet de l'amendement que je vous soumets. Il permettra de faciliter le recours au financement participatif par les collectivités territoriales, tout en maintenant une approche équilibrée, limitée aux champs pour lesquels ce financement peut être utilement mobilisé. Quel est l'avis de la commission des finances

une série de dispositions régissant les relations entre les autorités de régulation nationales et les commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un marché réglementé. En particulier, le règlement européen n° 537/2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public est venu préciser les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes doivent informer les autorités de régulation nationales. Outre le devoir d'information de l'Autorité des marchés financiers (AMF) par les commissaires aux comptes, en cas de refus de certifier les comptes ou de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, a introduit un devoir d'information à la charge des commissaires aux comptes, s'ils ont connaissance d'une information qui peut entraîner une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ; un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation ou un refus d'émettre un avis d'audit sur les états financiers ou l'émission d'un avis défavorable ou d'un avis assorti de réserves. Le droit français n'ayant pas été adapté sur ce point à la suite de l'entrée en vigueur du règlement européen susvisé, vise à mettre l'article L. 621-22 du code monétaire et financier en conformité avec la réglementation européenne. En outre, le règlement européen impose ces obligations d'information aux entités d'intérêt public et permet aux États membres d'exiger des informations supplémentaires. Par ailleurs, il est souhaitable, dans un souci de cohérence, que les nouvelles obligations précitées, mises à la charge des commissaires aux comptes, s'appliquent également aux commissaires aux comptes des sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation. Enfin, l'article L. 621-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction actuelle, impose un devoir d'information de l'AMF par les commissaires aux comptes en cas de mise en oeuvre de la procédure d'alerte. instaure le devoir d'information de l'AMF par les commissaires aux comptes des entités d'intérêt public en cas de risques ou de doutes sérieux concernant la continuité d'exploitation, le règlement européen n° 537/2014 ne distingue pas selon la forme sociale de l'entité d'intérêt public. En l'état, l'article L. 621-22 du code monétaire et financier n'est donc pas conforme au règlement européen. Le présent amendement vise donc à rendre cette disposition compatible avec le règlement européen, tel que nous le prévoyons dans ce projet de loi.

en l'espèce, l'Autorité des marchés financiers, de demander des informations aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, afin de mener à bien leurs actions de supervision, sans restriction particulière sur le type d'informations sollicitées. Or la rédaction actuelle de l'article L. 621-25 du code monétaire et financier autorise l'Autorité des marchés financiers à demander uniquement des informations sur l'application par les prestataires de services d'investissement, et donc des sociétés de gestion de portefeuille, de leurs règles de bonne conduite. Cette restriction est de nature à empêcher le lancement par l'Autorité des marchés financiers d'actions de supervision impliquant les commissaires aux comptes de sociétés de gestion de portefeuille, afin notamment de juger de la solidité financière des sociétés de gestion et d'anticiper d'éventuelles difficultés suffisamment en amont. Cet amendement vise donc à corriger cette sous-transposition en permettant à l'AMF de demander aux commissaires aux comptes de sociétés de gestion de portefeuille tout renseignement concernant l'application de ses obligations professionnelles, telles que définies par les dispositions législatives et réglementaires. Je rappelle que, en application de l'article L. 621-23 du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

sur les moyens qui devraient être mis à la disposition de l'autorité environnementale. Il est problématique de confier au seul préfet de région le soin de décider de l'opportunité de mener une évaluation et celui d'autoriser le

jour appelle la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances (projet n°